La séance est reprise. des transports, mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence dans notre tribune officielle

Il est accompagné de ministres-présidents et de membres du Bundesrat, notamment du président de la commission des questions de l'Union européenne. Cette visite est pour moi l'occasion de manifester l'attachement du Sénat à l'amitié franco-allemande et à son rôle irremplaçable au sein de l'Union européenne. Cette amitié, qui a été forgée après des siècles d'affrontements, a été scellée par le traité de l'Élysée, signé en 1963- nous avons en mémoire cette page de l'histoire -entre le général de Gaulle et le Chancelier Adenauer, et réaffirmée, le 22 janvier dernier, par le traité d'Aix-la-Chapelle, signé par la Chancelière Angela Merkel et le Président de la République française Emmanuel Macron. C'est grâce à la solidité du couple franco-allemand que nous avons réussi à construire une Europe qui symbolise la paix et la prospérité et à surmonter les crises. Nous ne devons pas l'oublier ! Aujourd'hui, face aux nombreux défis auxquels l'Europe est confrontée, la France et l'Allemagne doivent, plus que jamais, se montrer unies et raisonner en termes de communautés de destin. Comme en témoigne votre visite, le Sénat et le Bundesrat sont des acteurs engagés de cette relation. Je tiens d'ailleurs à saluer l'action de nos deux présidents de groupes d'amitié, Mme Catherine Troendlé et M. Tobias Hans, ainsi que les membres des deux groupes d'amitié, qui ne cessent de conforter l'amitié franco-allemande. Aujourd'hui, nous avons signé une déclaration commune, élaborée sur la base des travaux conduits par les présidents des commissions des affaires européennes de nos deux assemblées, nos collègues Guido Wolf et Jean Bizet, que je tiens à remercier. Cette déclaration commune traduit notre volonté de renforcer la coopération et les échanges entre le Sénat et le Bundesrat et de contribuer ainsi au nouvel élan qui doit être donné à la relation franco-allemande. entre le bicamérisme en Allemagne et en France, notamment en matière législative ou de contrôle de l'exécutif- sur cette question, nous ne renonçons naturellement nos deux assemblées partagent en effet un intérêt commun pour les questions européennes, pour la coopération décentralisée et transfrontalière et pour la subsidiarité, ce principe souvent méconnu dans notre pays, qui est pourtant gage de démocratie, de proximité et d'efficacité. Alors que l'Europe est trop souvent perçue comme éloignée des citoyens, j'ai la conviction que les parlements nationaux, et les chambres hautes en particulier, ont un rôle essentiel à jouer, notamment en tant que gardiens de la subsidiarité et pour lancer des initiatives communes, afin de rapprocher l'Europe des citoyens. Nous nous retrouverons du 13 au 15 juin à Paris, puisque nous recevrons ensemble les présidents des secondes chambres membres de l'Association des Sénats d'Europe. Nous rencontrerons à cette occasion les présidents de plusieurs Sénats du continent africain afin de dialoguer ensemble et d'apporter des réponses communes aux défis du développement, du climat, des migrations et de la paix.

Le général de Gaulle déclarait : « L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelles du peuple français et du peuple allemand.

Mes chers collègues, nous célébrons tout au long de cette semaine la francophonie, dont la Journée internationale se tiendra demain. Le drapeau de la francophonie et celui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que vous voyez dans notre hémicycle participent de cette célébration à laquelle s'associent les autres parlements des pays de la grande famille francophone. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, d'orientation des mobilités (projet n° 157 rectifié, texte

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a un an, je présentais le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Cette réforme répondait à une ambition forte : remettre sur pied notre système ferroviaire et lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle de colonne vertébrale de nos transports. C'était une étape essentielle dans la refonte de notre politique de mobilité voulue par le Président de la République et le Premier ministre ; je me souviens que le Sénat avait été au rendez-vous. ans après la LOTI, le projet de loi d'orientation des mobilités que j'ai l'honneur de présenter devant la Haute Assemblée est une deuxième étape. Les exigences de cette refondation n'ont pas changé exigence d'efficacité, d'abord, pour remettre en état notre système de transport aujourd'hui menacé par des décennies de sous-investissement exigence de justice sociale et territoriale, ensuite, afin qu'aucun de nos concitoyens, dans aucun de nos territoires, ne soit entravé dans sa mobilité et assigné à résidence exigence environnementale, enfin, avec la ferme volonté d'accélérer notre transition vers une mobilité plus durable, plus sobre et plus propre. Au terme du grand débat national, cette triple exigence résonne aujourd'hui avec une particulière acuité. Sur les ronds-points, dans les cahiers de doléances, au cours des réunions d'initiatives locales ou au travers des contributions se sont exprimées des colères, des attentes, des propositions. Ce sont celles auxquelles font face les élus locaux depuis des années. Ce sont celles que j'ai entendues dans le cadre du grand débat en Côte-d'Or, dans le Tarn, dans le Morbihan ou ailleurs, et je les partage. Ce sont celles d'une France à deux vitesses d'une France qui a offert toujours plus de vitesse aux uns et la galère de trains trop lents, trop bondés ou trop rares aux d'autres ; d'une France où il faut presque autant de temps pour rejoindre Bordeaux depuis Massas à seulement que depuis Paris par le TGV ; d'une France dans laquelle l'absence d'alternative à la voiture individuelle enferme celles et ceux qui sont trop jeunes, trop âgés ou qui n'ont tout simplement pas ou plus les moyens d'avoir une voiture. La crise des « gilets jaunes » a rappelé sans détour ce diagnostic, reflet des fractures sociales et territoriales qui minent notre pays depuis des décennies. Le projet de loi que je vous propose entend être une réponse structurelle à ces fractures. Il est le fruit d'un dialogue exigeant, constructif et sincère depuis bientôt deux ans avec les collectivités, les associations et les entreprises pour apporter des solutions concrètes et efficaces à chacun de nos concitoyens. Ce dialogue, engagé à l'occasion des Assises nationales de la mobilité, n'a eu de cesse de se poursuivre à chaque étape de la construction du texte. Au-delà de la méthode, qui me semble la bonne, ce dialogue était indispensable, car, en matière de mobilité, ce n'est pas l'État seul, et encore moins depuis Paris, qui est l'échelon compétent ou le plus pertinent. Ce n'est pas l'État qui conçoit des solutions avec des véhicules en libre-service à Charleville-Mézières et ses alentours, c'est Ardenne Métropole. Ce n'est pas l'État qui s'assure que les offres de mobilité à l'échelle de la Bretagne sont bien coordonnées, c'est la région. Ce n'est pas l'État qui propose la meilleure solution aux salariés d'une zone d'activité en Coeur de Beauce, c'est la communauté de communes en liaison avec les employeurs. C'est l'une des attentes qui s'est exprimée avec force dans le cadre du grand débat, à savoir plus de proximité dans les décisions et l'action publiques. Ce n'est pas pour autant moins d'État qui nous est demandé et que je vous propose, car son rôle est fondamental dans cette nouvelle architecture. Il revient à l'État de fixer un cap clair à l'État de donner les outils et les moyens pour apporter les meilleures réponses au meilleur niveau ; à l'État de lever les freins pour libérer l'innovation ; à l'État de rendre crédibles ses engagements. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet de loi que je vous propose. Dans ce contexte, la première mission du législateur est de veiller à ce qu'il y ait à chaque niveau un interlocuteur identifié. Aujourd'hui, il existe des « zones blanches » de la mobilité. Cette faille structurelle a des conséquences très directes pour nos concitoyens. Dans 80 % du territoire, il n'y a pas de solution proposée par une autorité organisatrice « dédiée » à la mobilité. Cette situation n'est plus acceptable. C'est pourquoi la loi a pour objectif prioritaire de simplifier l'exercice de la compétence mobilité par les collectivités, notamment par les communautés de communes, afin que celles-ci puissent mettre en place des solutions de proximité, simples et adaptées aux besoins. La commission a souhaité ajouter un délai de six mois pour cette prise de compétence. Je n'y suis pas opposée, dès lors que les collectivités concernées sont d'accord. En effet, je rappelle que les mesures contenues dans le volet « gouvernance » ont toutes été prises en étroite concertation avec les collectivités et leurs associations. Il me semble donc important de maintenir les grands équilibres trouvés dans la concertation. Le bon niveau de réponse aux questions de mobilité, c'est le bassin de mobilité, avec un rôle de coordination de la région. Vous avez proposé la mise en place de contrats opérationnels de mobilité et le renforcement de la concertation entre la région et les collectivités. J'y suis bien évidemment favorable, puisque c'est la même logique qui soutient la création du comité des partenaires pour associer les usagers et les employeurs à la définition des offres. Répondre au plus près des besoins, c'est aussi se donner les moyens d'apporter des réponses spécifiques à nos concitoyens les plus fragiles. Le projet de loi prévoit donc la possibilité, pour les autorités organisatrices, d'apporter des aides et des services spécifiques à ces publics, avec un souci de coordination avec tous les acteurs qui les accompagnent. C'est dans cette logique que je vous propose la mise en place de plans d'action communs en faveur de la mobilité solidaire, élaborés à l'échelle d'un bassin de mobilité, pour permettre à chacun d'accéder plus facilement à l'emploi, à la formation ou aux services publics. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai eu l'occasion de le dire, ce projet de loi est une boîte à outils, pensée avec et pour les collectivités ainsi que tous les acteurs de la mobilité.

Une boîte à outils, cela veut dire que l'on facilite et que l'on aide financièrement les élus qui veulent mettre en place des solutions de covoiturage, des véhicules électriques en libre-service ou du transport à la demande. d'ores et déjà prévu de mobiliser 500 millions d'euros durant le quinquennat au travers de la dotation de soutien à l'investissement local, pour soutenir financièrement ce type de projets concrets. Cela n'est pas assez connu, et j'invite les élus à s'en saisir dans les territoires, en liaison avec les préfets l'État est bien là. Pour apporter les meilleures réponses à la diversité des besoins, nous pouvons compter sur le formidable potentiel offert par l'innovation. La loi portera l'ouverture des données en temps réel des offres de mobilité pour voir émerger de nouveaux services porte-à-porte. Autre élément essentiel : l'accès aux services de vente. C'est la condition nécessaire à l'émergence de services intégrés de mobilité. Nous devons encore trouver un bon équilibre entre la mission des autorités organisatrices et les initiatives des acteurs économiques. La loi donnera également tous les outils nécessaires pour accompagner le développement de l'autopartage, le transport à la demande ou le covoiturage, avec de nouveaux leviers, en vue de permettre leur déploiement ou encore, très prochainement, la mise en service de navettes autonomes. Ces innovations ne doivent pas être l'apanage des grandes villes, mais elles doivent profiter à tous dans tous les territoires. La méthode à laquelle je crois, c'est un cadre normatif adapté et une impulsion. C'est tout l'objet de la démarche France Mobilités : elle permet le développement et la diffusion de ces innovations par l'accompagnement et la mise en relation des territoires et des porteurs de solutions. Les projets soutenus sont d'une remarquable diversité. Je vous invite d'ailleurs à relayer les soixante-dix projets nés dans vos territoires, car ils sont une illustration opérationnelle de cette « intelligence des territoires » à laquelle le Sénat est, je le sais, attaché. Je lancerai prochainement une plateforme en ligne, France Mobilités, pour mieux les faire connaître. Ne soyons pas naïfs ! Ces innovations posent aussi un certain nombre de défis, qui nécessitent une régulation adaptée. Je pense notamment aux nouveaux services de mobilités en libre-service et au nécessaire cadre de protection pour les travailleurs de cette nouvelle économie. Ce sont des sujets importants, et nous aurons à en débattre. Ne soyons pas non plus attentistes ! Nous devons avoir en permanence un temps d'avance. C'est pourquoi nous proposons une habilitation portant sur l'expérimentation dans le monde rural. Celle-ci permettra d'avoir un cadre pour imaginer et tester de nouveaux services entre particuliers en expérimentant, par exemple, l'assouplissement de certaines règles liées au covoiturage, sans prendre le risque de créer une concurrence déloyale vis-à-vis des professionnels. un mot sur les ordonnances. Je sais que les commissions se sont émues du nombre d'ordonnances. Les rapporteurs pourront en témoigner, nous avons partagé les textes qui étaient d'ores et déjà disponibles. Le choix de passer par ordonnances s'explique principalement par le niveau de technicité, qui aurait eu pour conséquence d'alourdir considérablement la loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons prendre une autre révolution à bras-le-corps, celle de la transition écologique elle est une chance, pour que nous changions durablement notre façon de nous déplacer. Le projet de loi s'inscrit dans l'agenda ambitieux de l'accord de Paris et du plan Climat. Il fixe des objectifs clairs, progressifs, partagés, qui permettent à tous d'anticiper et d'être acteurs de la transition. Il prévoit des mesures d'accompagnement concrètes afin que cette transition ne laisse personne sur le bord de la route. Des transports plus économes, c'est un impératif pour la planète, c'est aussi une opportunité pour nos concitoyens. C'est en ce sens que nous proposons des dispositifs de soutien aux usages vertueux. Je pense au « forfait mobilités durables » pour permettre aux employeurs de soutenir le covoiturage et le vélo. Je pense aussi à la conversion des parcs, avec, notamment, la prime à la conversion ou le soutien au déploiement des infrastructures de recharge et d'avitaillement. Je vous propose aussi des mesures fortes pour développer les mobilités actives. Je suis heureuse de voir que l'impulsion du plan Vélo a bien été relayée par votre commission, avec des apports nécessitant peut-être quelques ajustements, mais ceux-ci vont dans le bon sens. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, ce texte a pour ambition d'apporter des réponses au plus près des besoins. Cela rejoint pleinement ce qui s'est exprimé dans le grand débat, dont je tire trois enseignements. enseignement : nos concitoyens ont besoin de solutions « sur mesure ». Aussi, nous travaillons avec Muriel Pénicaud, Jacqueline Gourault, les partenaires sociaux et les associations d'élus pour renforcer le « forfait mobilités Les discussions avancent, et je souhaite que nous aboutissions dans les prochaines semaines, afin de rendre ce forfait systématique, voire obligatoire. De la même façon, la prime à la conversion doit être complétée. Pour certains de nos concitoyens, le reste à charge est encore trop élevé et ne permet pas de franchir le pas. Je suis favorable à des solutions de microcrédits ou de location longue durée ; nous y travaillons avec ma collègue Christelle Dubos. Deuxième enseignement : la proximité et la subsidiarité. Plus personne ne comprend que les décisions doivent systématiquement remonter à Paris. Tel est bien l'esprit du projet de loi. Aussi, je vous propose d'aller plus loin sur un sujet qui vous est cher, celui des petites lignes ferroviaires. Ces lignes, qui n'ont de « petites » que le nom, ont été les grandes sacrifiées de notre réseau ferroviaire pendant des décennies elles accusent aujourd'hui un retard en termes d'investissement, que nous devons rattraper. Avec la réforme ferroviaire, nous avons engagé un effort sans précédent dans la régénération du réseau et nous avons confirmé les engagements de l'État dans les contrats de plan État-région. Mais nous devons faire mieux, en engageant un plan de bataille région par région pour redonner un avenir aux petites lignes. Sans attendre les conclusions de la mission que j'ai confiée au préfet Philizot, j'ai souhaité répondre à la demande exprimée par plusieurs régions de gérer directement certaines de ces lignes. Pourquoi s'y opposer au moment où le pays aspire à davantage de proximité ? Tel est le sens de l'amendement que le Gouvernement a déposé. Ce que je retiens aussi des attentes exprimées par les territoires, c'est la nécessité de recréer de la confiance dans la parole publique et, plus particulièrement, dans les engagements de l'État. Telle est l'ambition de la programmation des infrastructures. Cette programmation, c'est d'abord le fruit d'un travail exigeant et reconnu, celui du Conseil d'orientation des infrastructures, dont je veux de nouveau saluer ici les membres siégeant ou ayant siégé sur ces travées : le président Maurey, le sénateur Dagbert et votre ancien collègue Gérard Cornu. Cette programmation, c'est également le fruit de choix difficiles et assumés pour mettre fin à des décennies de promesses non tenues ; j'ai déjà eu l'occasion de les présenter dans cet hémicycle lors des débats que vous avez utilement engagés. Votre commission a fait le choix d'en faire le premier titre de la loi. Je le déplore, car je considère que cette première place revient aux collectivités, qui seront, demain, les plus à même d'apporter les solutions concrètes que nos concitoyens attendent.

Cette programmation, c'est une forte augmentation des investissements de l'État, avec 13,4 milliards d'euros sur cinq ans, soit 40 % de plus qu'au cours du dernier quinquennat. est le contraire d'une liste de grands projets. Elle consacre la priorité donnée aux transports du quotidien avec cinq grands programmes prioritaires : l'entretien et la modernisation des réseaux existants ; la désaturation des grands noeuds ferroviaires ; l'accélération du désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux le développement de l'usage des mobilités propres, partagées et actives ; le soutien au report modal dans le transport de marchandises. Au sein des grands projets, priorité est donnée aux opérations concourant d'abord à l'amélioration des déplacements du quotidien. Le choix et le calendrier des projets qui seront financés ont été pris en concertation et sont cohérents. Je ne peux donc que vous mettre en garde contre la tentation d'ajouter tel ou tel projet à la liste, sans conserver la cohérence des enveloppes globales. Cette programmation, c'est un cap clair que je vous propose de partager, une vision sur dix ans, déclinée en priorités. J'ai entendu, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, les interrogations, voire les inquiétudes concernant le financement de cette programmation et, plus largement, de ce texte je veux y répondre. Sur la forme, tout d'abord : vous le savez, les financements n'ont pas vocation à figurer dans cette loi, car il ne s'agit pas d'une loi de finances. En cela, ce projet de loi ne diffère pas des autres exercices de programmation auxquels vous êtes habitués. Je pense à la loi de programmation militaire que vous avez adoptée.

2020 et les années suivantes, la question du financement reste en débat. Vous le savez, nous aurons à dégager 500 millions d'euros supplémentaires par an à partir de l'an prochain. Sur ce sujet, qui, je le sais, suscite beaucoup d'intérêt, nombre de nos concitoyens ne comprennent pas que des files de camions traversent notre pays sans faire le plein en France et donc sans contribuer au financement de nos infrastructures. C'est un sentiment que je partage, et leur contribution me paraît être une piste légitime. Mais nous n'arrêterons aucune décision en la matière avant d'avoir étudié toutes les propositions issues du grand débat. la question des ressources disponibles pour les collectivités ne mettant pas en oeuvre des services réguliers ou dont le potentiel fiscal est insuffisant. Votre commission a fait le choix d'introduire dans ce texte des dispositifs de financement. Cela me semble prématuré, car de nombreuses questions sont ouvertes. Le versement mobilité à 0,3 %, introduit en commission, est un prélèvement complexe à mettre en oeuvre ; ce n'est peut-être pas la meilleure réponse. D'autres options sont possibles, je pense notamment à la CFE. De même, nous devons continuer à travailler sur les mécanismes de solidarité pour les collectivités les plus fragiles. Mais je veux l'exprimer clairement devant vous : pas de prise de compétence sans ressources adaptées. Dans les deux cas, il y a donc un engagement du Gouvernement à trouver des réponses qui auront leur place dans la réforme de la fiscalité locale. Surtout, et sans attendre ces échéances, l'État mobilise d'ores et déjà de nombreux leviers pour accompagner les initiatives locales, qu'il s'agisse des appels à projets de l'Ademe, des certificats d'économies d'énergie- 60 millions d'euros ont été mobilisés en faveur du vélo au cours des derniers mois -ou encore, comme je l'ai déjà évoqué, de la dotation de soutien à l'investissement local, à hauteur de 100 millions d'euros par an. Nous aurons ce débat, mesdames, messieurs les sénateurs, et je m'en réjouis. Avant de conclure, je voudrais signaler que le projet de loi comporte des dispositions sur le cadre social pour accompagner l'ouverture à la concurrence des transports urbains franciliens, votée voilà dix ans. À l'issue d'une cinquantaine de réunions de concertation menées avec les organisations syndicales représentatives, dont je tiens à souligner l'esprit de responsabilité, les employeurs et, naturellement, l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilités, le Gouvernement a déposé une série d'amendements visant à préciser les garanties sociales conservées par les salariés de la RATP en cas de transfert. Mesdames, messieurs les sénateurs, votre regard et l'expérience qui est la vôtre des collectivités locales seront précieux pour enrichir ce texte. Je mesure le travail accompli en commission, et je me réjouis que l'équilibre général du texte en sorte conforté. Je souhaite remercier le rapporteur pour la qualité des échanges que nous avons eus et l'approche constructive qu'il a adoptée, avec le soutien de l'ensemble des membres de la commission et du rapporteur pour avis. Vous l'aurez compris, ce projet de loi, construit dans la concertation, s'adresse en premier lieu aux territoires et a pour vocation de répondre aux grands enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain, au service de tous et de tous les territoires. Il est de notre devoir à tous de répondre à cette fracture territoriale et sociale, devenue insupportable pour nos concitoyens. Les ambitions sont claires et, je crois, partagées. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous allons examiner durant les deux prochaines semaines est très attendu. Depuis la fin des Assises nationales de la mobilité en 2017, les acteurs de la mobilité appellent au développement de nouvelles offres de transports. Les collectivités territoriales attendent, elles, une meilleure gouvernance et une sécurisation de ce développement. Surtout, de très nombreux Français réclament de vrais changements. Ils sont des millions Ce sont ceux qui vivent dans ce que vous appelez à juste titre, madame la ministre, les « zones blanches de la mobilité »- on les nomme aussi les « assignés à résidence ». Ce sont ceux qui vivent au quotidien les inégalités en matière de transport, condamnés à prendre leur voiture pour aller travailler, faute de moyens ou d'alternatives existantes. Ces Français subissent aujourd'hui une « double peine », puisqu'ils paient à la pompe des taxes qui ne servent même plus à financer la remise en état de nos routes et le développement d'alternatives à la voiture individuelle. Ils ont moins de moyens, moins de choix et ils payent toujours plus l'un des éléments déclencheurs de la crise qui n'en finit pas de secouer notre pays. L'équation est simple à énoncer, mais difficile à résoudre : comment faire pour que la révolution des mobilités soit, non pas une machine de plus à créer des gagnants et des perdants, mais, au contraire, une machine à « désenclaver » Un grand nombre de mesures de votre projet de loi vont dans le bon sens : meilleure gouvernance, soutien au développement des mobilités propres, plus grande sécurité dans nos réseaux de transport. Les acteurs que nous avons rencontrés nous ont tous dit qu'ils avaient été largement associés à la construction de texte, même si beaucoup de sujets ont disparu au fil des arbitrages successifs de Bercy et de Matignon. Mais, au-delà de ces avancées, subsiste malheureusement une faiblesse majeure qui compromet l'efficacité des mesures proposées : je parle évidemment de l'absence de moyens à la hauteur des enjeux. Certes, comme vous le répétez souvent, ce projet de loi n'est pas un projet de loi de finances et, effectivement, on peut le voir comme une boîte à outils. Mais combien de sujets ont été renvoyés, au cours des derniers mois, à l'examen de ce texte ? Et comment pourrait-on passer sous silence les 28 milliards d'euros d'investissement de l'État prévus dans le secteur des transports pour les dix prochaines années ? Vous demandez aujourd'hui à notre assemblée de voter une trajectoire financière de dépenses, alors que les ressources prévues ne sont ni suffisantes, ni stabilisées, ni même, pour certaines, encore connues. il apparaît clairement que cette programmation suppose, non seulement une ressource complémentaire, que vous estimez à 500 millions d'euros, mais également un niveau de recettes provenant des amendes radars défiant toute crédibilité, afin de compenser la baisse prévisionnelle annoncée de la part des taxes sur les carburants affectée au financement des infrastructures, qui devrait chuter de 1,1 milliard d'euros, à 526 millions d'euros en 2022. Face à ce constat, et avec le peu de marges de manoeuvre dont nous disposons, notre commission a fait des choix clairs. Elle souhaiterait que vous puissiez les entendre, afin de garantir la soutenabilité de la programmation. Tout d'abord, elle n'a pas cédé à la facilité consistant à augmenter artificiellement les dépenses de tel ou tel programme d'investissement ou de telle ou telle priorité. Alors même que le niveau de dépenses que vous avez retenu se situe bien en deçà du scénario central préconisé par le Conseil d'orientation des infrastructures, lequel impliquait 3 milliards d'euros d'investissement par an, la commission a préféré garantir le financement de cette trajectoire, fût-elle décevante, plutôt que de tomber dans les écueils des programmations précédentes et renoncer à toute crédibilité. Nous avons également sanctuarisé les ressources de l'Afitf, afin d'asseoir la programmation sur des recettes crédibles.

garantirait un niveau de TICPE affectée au financement de nos infrastructures de 1,2 milliard d'euros par an. Il s'agit d'une mesure de justice, qui s'inscrit dans la perspective d'une fiscalité écologique acceptée. N'oublions pas que, en 2014, lorsque nous avons taxé les Français qui prennent leur voiture pour aller travailler et les poids lourds, c'était pour financer nos infrastructures ; or cet argent a progressivement été détourné vers le budget général, comme dans bien d'autres cas, d'ailleurs ! Comment aujourd'hui demander à nouveau 500 millions d'euros L'économiste Jean Pisani-Ferry lui-même, artisan du programme économique de campagne du Président de la République, a reconnu très récemment dans une tribune le caractère régressif de la taxe carbone, qui s'est traduite par une perte importante de pouvoir d'achat, non compensée pour les classes moyennes et populaires. Pour lui, la leçon est claire : « Pour que la taxe carbone soit acceptée, il ne faut pas qu'elle rapporte à l'État. » Le produit doit en effet être intégralement redistribué pour la transition écologique et la compensation des pertes de pouvoir d'achat. Il ajoute même : « Chaque euro prélevé doit être rendu. » Cette règle nous semble juste. C'est le choix que fait notre commission : affectons à la transition écologique dans le domaine des transports les taxes que nous prélevons déjà sur les carburants. Sur les 17 milliards d'euros de TICPE prélevés par l'État, une somme allant de 1,6 milliard à 1,8 milliard d'euros devrait, selon nous, être fléchée vers l'entretien de nos routes et la régénération de nos réseaux. représente le produit de l'augmentation de 2014, auquel il conviendrait d'ajouter, en moyenne, entre 400 millions et 600 millions d'euros dans les années à venir pour garantir la soutenabilité de votre programmation, sur la route comme sur le rail ou pour d'autres moyens de transport. Ce principe simple permet un financement à la hauteur des ambitions.

Le manque de transparence sur l'affectation de la fiscalité écologique a été l'un des facteurs déclencheurs du mouvement des « gilets jaunes ». Nous avons donc souhaité prévoir un volet dédié au contrôle de la programmation.

brièvement le choix de notre commission de ne pas faire figurer la liste des projets d'infrastructures dans le corps du projet de loi ou du rapport annexé, afin de respecter une logique de moyens, plutôt que de céder à la tentation de promesses non financées. Nos collègues, nombreux, qui ont déposé des amendements pour inscrire tel ou tel projet doivent néanmoins pouvoir interpeller le Gouvernement et obtenir des réponses au cours du débat. La commission, attentive à leurs préoccupations, a introduit deux dispositifs importants la réévaluation quinquennale des projets sous l'égide du COI et l'inscription, dans le rapport annexé, de l'objectif de répondre à terme aux calendriers ambitieux prévus par le scénario 3 établi par le Conseil. Avec cette double garantie, la commission demandera aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. » du projet de loi, notre commission a donné aux collectivités, notamment les plus rurales, les moyens que la rédaction du Gouvernement ne prévoyait pas pour organiser les services de mobilité : une extension du versement mobilité aux collectivités n'organisant pas de services réguliers l'attribution d'une partie du produit de la TICPE aux territoires ruraux dont les ressources seraient insuffisantes ; le fléchage des certificats d'économies d'énergie vers la mobilité propre. Madame la ministre, vous avez déposé des amendements de suppression afin de revenir sur ces avancées, mais sans rien proposer en échange. Je ne vous le cache pas, la balle était pourtant dans votre camp ! Nous aurions été prêts à envisager d'amender, pour améliorer ces dispositifs En matière de gouvernance, notre commission a apporté souplesse et sécurité pour les acteurs, au premier rang desquels les collectivités territoriales. Elle a notamment allongé le délai accordé aux communes pour décider du transfert de la compétence d'organisation des mobilités aux communautés de communes, ainsi que celui dont disposent les autorités organisatrices de la mobilité pour élaborer leur plan de mobilité. Elle a également prévu un nouveau cas de réversibilité pour les communautés de communes souhaitant récupérer la compétence, en commun accord avec la région. Je tiens à préciser que cette réversibilité ne sera pas possible sans l'accord express des régions- c'est important

Concernant les nouvelles mobilités, le développement rapide des services de pose un certain nombre de difficultés, notamment en termes de régulation, de sécurité et de tranquillité publiques. Notre commission a adopté un amendement renforçant les pouvoirs des autorités organisatrices,

le développement de ces nouveaux services. Là encore, madame la ministre, vous nous proposez de revenir à votre texte initial. Tout en reconnaissant ses faiblesses, vous ne proposez aucune alternative. La commission a également adopté de nombreux dispositifs permettant d'améliorer les offres de mobilité dans les zones peu denses, au travers du renforcement du « forfait mobilités durables » ou encore d'une meilleure modulation du tarif de raccordement aux infrastructures de recharge publique. Elle a considérablement renforcé le volet dédié aux modes de transports peu polluants, ainsi que celui qui a trait à la sécurité routière et à la sûreté dans les transports.

été nombreux à déposer des amendements, tombés en commission sous le coup de l'article 40. Nous avions exprimé fortement le souhait que vous puissiez nous présenter un dispositif en séance sur cette question importante. C'est chose faite, et je suis heureux que le Sénat puisse en débattre en toute transparence, plutôt que d'en passer par des ordonnances plus techniques. Mes chers collègues, pour conclure, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous, en particulier les membres de la commission de l'aménagement du territoire et leur coopération et leur attitude constructive tout au long de nos travaux et de la centaine d'auditions que nous avons menées. Je remercie Mme la ministre pour la qualité et la régularité des échanges que nous avons pu avoir, le président de la commission Hervé Maurey, Françoise Gatel, rapporteur pour avis de la commission des lois,

européennes. Je suis convaincu que nous aurons des débats riches et de qualité, car nous partageons tous le même objectif : en finir, une bonne fois pour toutes, avec les fractures territoriales. La parole

Ce projet de loi s'inscrit dans une actualité sociale très lourde, née d'un sentiment de déclassement fort et qui a explosé, si je puis dire, à l'occasion d'une augmentation du coût du carburant, en novembre Le défi de la mobilité se double d'une formidable opportunité liée aux innovations, qui créent un bouleversement inédit depuis l'émergence de la voiture individuelle. La commission des lois a fait le choix de se concentrer sur les dispositions relevant strictement de sa compétence, laissant à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable l'initiative de se prononcer sur les autres sujets. La saisine de la commission des lois concernait donc 16 articles, couvrant cinq thématiques : la définition et la répartition des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, la protection des données personnelles, la sécurité routière, le droit pénal et la sûreté dans les transports, la domanialité et la commande publiques. Ce sont 24 amendements qui ont été proposés et adoptés par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, visant à mieux adapter le texte aux réalités locales, à apporter une plus grande sécurité juridique et à garantir la proportionnalité de certaines dispositions. Le premier axe de la commission des lois a été de favoriser l'exercice des compétences de mobilité par les collectivités territoriales. Nous avons sur ce point souhaité rappeler à tous l'architecture territoriale de notre pays et notre philosophie de l'intercommunalité. Les EPCI ne sont compétents que parce qu'ils se sont vu transférer la compétence par leurs communes membres. Sur le territoire des communautés de communes, le projet de loi prévoyait un mécanisme complexe pour favoriser la prise de la compétence d'organisation des mobilités par le niveau de collectivité le plus pertinent : l'intercommunalité ou la région. Notre commission a émis deux au 1 juillet 2021 l'échéance du transfert de la compétence aux régions par les communautés de communes qui le souhaiteraient, car, au vu des échéances électorales de mars 2020, la date initialement proposée ne permettait pas de garantir une prise de compétence sereine et pertinente. nous avons voulu ajouter, aux cas dans lesquels la communauté de communes peut demander à la région de reprendre la compétence d'organisation de la mobilité, celui d'un accord entre ces deux entités. Enfin, nous avons proposé plusieurs amendements pour améliorer et renforcer la coordination entre les différentes AOM, notamment dans la définition des bassins de mobilité. Sur cette première partie du projet de loi, le texte issu de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable semble équilibré. Je salue, plus particulièrement, l'introduction de différentes solutions de financement des services de mobilité. En effet, madame la ministre, l'intelligence de votre projet ne pouvait masquer son indigence financière. Pour protéger les données personnelles dans le domaine de la circulation des véhicules routiers, nous avons proposé de supprimer les habilitations que vous souhaitiez relatives aux traitements de données des « véhicules connectés ». Le champ nous paraissait large et imprécis,

certaines phases du traitement des données, nombreuses et très sensibles, ainsi captées, en prévoyant un masquage irréversible des photographies des passagers et des tiers. Par ailleurs, nous avons veillé à garantir l'équilibre et la proportionnalité des mesures de sûreté et de sécurité, en réservant à l'autorité judiciaire le soin de sanctionner les agressions contre les examinateurs du permis de conduire ; en garantissant la proportionnalité de certaines mesures, notamment en cas de non-paiement de péages sur autoroutes en encadrant mieux la possibilité ouverte aux exploitants de services de transport public de recourir à des équipes privées cynotechniques pour la détection d'explosifs

je souhaite saluer le rapporteur au fond, M. Didier Mandelli, dont les qualités d'écoute ont permis un véritable travail en commun. Le texte proposé nous satisfait sur les points dont la commission des lois s'était saisie pour avis. Madame la ministre, il appartiendra maintenant à l'État

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous allons examiner est centré sur les transports, plus particulièrement sur les transports humains

La politique européenne des transports entend faciliter les déplacements. Elle organise la coordination et la connectivité des différents modes de transport. Elle définit des exigences de sécurité. Enfin, elle comporte une dimension environnementale forte, avec des objectifs en matière de performance énergétique. Le paquet mobilité, en cours d'adoption, poursuit l'harmonisation et renforce toutes ces dimensions. Ainsi qu'elle l'a fait à quatre reprises depuis février 2018, la commission des affaires européennes a examiné le présent projet de loi dans le cadre de la mission de veille que lui a confiée la conférence des présidents, afin d'identifier d'éventuelles sur-transpositions du droit européen. Dès lors qu'une norme européenne s'impose dans tout État membre, il n'y a pas lieu d'y ajouter des contraintes nationales, sauf si celles-ci sont dûment justifiées. Il y va d'une bonne lisibilité pour nos concitoyens, du renforcement de leur sentiment d'appartenance à l'Union européenne et de la compétitivité de nos opérateurs économiques. Le projet de loi prévoit des mesures d'application de plusieurs règlements européens. Or, qui dit règlement, dit, en principe, peu de marges de manoeuvre, sous réserve des options qu'il ouvre. Quelques articles exploitent de telles options, sans ajouter au texte européen. C'est le cas de l'article 23, en matière de pré-équipement des parcs de stationnement pour l'installation de bornes de recharge des véhicules électriques, qui reprend la dispense en faveur des PME. L'article 9 va toutefois au-delà des obligations imposées par le règlement délégué, tout en s'inscrivant dans la logique de celui-ci. En effet, il prévoit l'ouverture, non seulement des données statiques de transports, mais également des données dynamiques, qui permettent de connaître l'état du trafic en temps réel. L'inclusion de ces données n'est pas une obligation, mais le règlement européen l'évoque dans un considérant et l'encadre dans son annexe. Le projet de loi semble également aller un peu plus loin que ne l'exigent les textes européens en matière de sanction du non-respect des limites d'émission de CO2 et de particules par différents engins. Mais, madame la ministre, le dispositif est renvoyé à des ordonnances Pour le reste, le projet de loi ne comporte pas de dispositions pouvant être qualifiées de sur-transpositions, sous réserve de mesures facilitant les déplacements des personnes à mobilité réduite- qui pourrait s'en insurger deux remarques pour conclure. Premièrement, plusieurs dispositions autorisent l'accès à des données à caractère personnel, notamment pour la surveillance des véhicules routiers connectés. Il convient de veiller strictement au respect du règlement général sur la protection des données et de la directive dite ePrivacy. cinq articles sont repris du projet de loi portant suppression de sur-transpositions, adopté par le Sénat en novembre dernier. Ils exploitent, pour l'essentiel, des dérogations ouvertes par la directive ferroviaire de 2012.

loi fondatrice de l'existence d'un droit au transport comme corollaire d'un service public. C'est un projet ambitieux ! Nous partageons l'idée d'une nécessaire redéfinition des besoins, pour créer les outils permettant de répondre aux enjeux nouveaux de déplacement, d'aménagement du territoire, de développement des technologies et, surtout, aux enjeux environnementaux, qui doivent nous conduire à la sobriété énergétique. La planète et nos concitoyens ne peuvent plus supporter cette pollution massive et continue, liée à l'activité humaine et aux flux mondiaux. Alors que les courbes des émissions de gaz à effet de serre, contrairement aux engagements de l'accord de Paris, sont reparties à la hausse, notre système de transport doit être compatible avec la lutte engagée contre le changement climatique. C'est bien l'« affaire du siècle Pourtant, ces enjeux sont mal traités dans le projet de loi. L'exigence du report modal, notamment pour le transport de marchandises, est sous-estimée ; la place du ferroviaire, comme du fluvial, mineure. Ce projet de loi, au fond, poursuit la voie engagée au cours des trente dernières années, ne proposant comme solution d'avenir que la libéralisation, le démantèlement des opérateurs publics et le désengagement de l'État, laissant une part prépondérante aux intérêts privés pour satisfaire l'intérêt général. une loi bien dans son temps qui, sous couvert de modernité, consacre la primauté des solutions individuelles sur le collectif. Or, faut-il le rappeler, l'addition de transports individuels n'a jamais fait un transport collectif. une loi qui manque de structure puisque, si elle traite bien les mobilités des trajets courts, elle passe totalement à côté de la nécessité de conserver la colonne vertébrale du système de transport que constituent les lignes ferroviaires, y compris des lignes de vie. une loi qui exclut, encore une fois, d'appréhender dans un même mouvement les questions de transports, de logements, d'emploi et de service public, alors même que l'éloignement de l'habitat des lieux de travail, le logement cher et l'étalement urbain sont à l'origine de l'allongement des temps de transport et induisent la saturation et l'engorgement des routes. Avec ce texte, nous travaillons donc, non pas sur les causes de l'accroissement du besoin de mobilité, mais sur les modalités de réponse à ce besoin, ce qui nous paraît constituer une lacune importante. quelques remarques sur la forme- comme souvent, elles rejoignent le fond. Nous sommes particulièrement inquiets du recours inédit sur ce texte, pour l'étude d'impact et l'exposé des motifs, aux services d'un cabinet privé, comme si les compétences n'existaient pas en interne. Ce choix n'est pas un hasard. laisse le soin à d'autres de définir l'intérêt public nous préoccupe, notamment quand cela touche à des actes aussi régaliens que la rédaction d'un projet de loi. Plus grave encore, alors que le Gouvernement s'était engagé à repousser l'examen du texte à l'issue du grand débat, il n'en est rien. Pourtant,

du coût du transport, mais aussi celle des conditions d'un égal accès de tous à l'emploi, au service public, à la santé, à la culture ... En effet, nous le savons tous, le droit au transport conditionne concrètement l'exercice d'autres droits. Nous aurions donc souhaité que ce projet de loi tienne compte des aspirations de nos concitoyens et considérons que son examen, dans cette enceinte, est prématuré. Sur le fond, il s'agit d'un texte fourre-tout- vous le qualifiez vous-même, madame la ministre, de boîte à outils abordant pêle-mêle le covoiturage, les trottinettes, le vélo, le bus ... sans aucune cohérence. Inversement, nous voyons dans le cadencement des réformes une grande cohérence. L'année dernière, avec la réforme ferroviaire, vous avez enterré le train. Nous pouvons donc aujourd'hui parler des autres mobilités : « Vous n'avez plus de train, prenez votre trottinette ou optez pour le covoiturage ! » Telle est la philosophie de ce projet de loi, qui renvoie la définition de l'offre de transport à chaque autorité organisatrice, selon ses moyens, des intercommunalités aux régions, laissant craindre de grandes inégalités territoriales et une balkanisation de l'offre de transport. Le changement sémantique illustre parfaitement cette stratégie. Nous ne parlerons donc plus du « droit au transport », droit fondé sur un maillage territorial, une offre structurante de masse, mais du « droit à la mobilité », aux contours flous et à la définition évanescente, laissant les individus libres de choisir leur mobilité, comme si l'offre de transports n'était pas directement le résultat de l'investissement public et de choix politiques. Ce changement terminologique s'explique par le passage d'un système de transport public, opéré par des opérateurs publics, publics, à des solutions individuelles ou reposant sur l'initiative privée, des solutions qui ont d'ailleurs toutes pour point commun d'emprunter la route. L'avenir de la route, c'est donc ... la route Bel effort pour la transition écologique ! Bien sûr, nous ne sommes pas opposés au développement du vélo, de la marche ou d'autres mobilités décarbonées, mais nous voulons aussi aborder la question du service public, des transports collectifs et d'une politique publique. Nous voulons également aborder la question des financements, grande inconnue de ce projet de loi. Le Gouvernement fait le choix du scénario 2 du COI, ce qui nous paraît faible. Pire encore, malgré les annonces d'un effort de 40 % de financements supplémentaires, c'est le silence radio sur les financements nouveaux pour l'Afitf. Soulignons tout de même les efforts évidents et remarquables du rapporteur, qui a permis- c'est déjà bien -de sanctuariser la part de la hausse de la TICPE attribuée à l'Afitf et d'attribuer une nouvelle portion de cette recette aux collectivités. Des efforts de fléchage, donc, mais pas de sources nouvelles ! Nous y reviendrons par nos amendements, en proposant des financements nouveaux, à la fois pour les autorités organisatrices au travers du versement transport ou de la baisse de la TVA et pour l'Afitf. Nous proposerons ainsi la mise en oeuvre d'une taxe poids lourds : il faut bien revenir sur cet avantage concurrentiel de la route, qui ne finance pas les infrastructures. Parce qu'il s'agit aussi de justice et d'efficacité fiscales, nous pensons que les exonérations fiscales des camions seraient mieux employées pour le financement de l'Afitf, tout comme nous considérons que l'État aurait intérêt à retrouver la maîtrise de ses infrastructures, au premier chef des concessions autoroutières, ou, pour le moins, à ne pas en autoriser de nouvelles, comme le fait ce projet de loi. L'État doit reprendre la main Enfin- c'est le troisième argument, et non le moindre, qui justifie cette motion de procédure, nous sommes farouchement opposés à la libéralisation des transports urbains et à l'explosion de la RATP en une myriade de filiales au gré des contrats obtenus. Nous considérons que l'organisation de la filialisation correspond de la filialisation correspond à une stratégie connue : segmenter pour mieux privatiser ensuite les opérateurs publics. Certes, cette ouverture à la concurrence est prévue depuis l'adoption du règlement OSP et de la loi de 2009. Certes, les possibilités de dérogation pour le transport urbain n'existent pas dans ce règlement, contrairement au ferroviaire. Mais nous continuons de penser que cet horizon n'est pas indépassable, y compris parce qu'il va s'avérer coûteux pour les autorités organisatrices dans l'organisation des procédures. Nous considérons, à l'instar de ce que nous avons soutenu l'année passée pendant la réforme ferroviaire, que la France s'honorerait à porter au niveau européen l'exigence d'une révision des traités et des directives qui imposent la concurrence en tout domaine. Nous avons l'expérience aujourd'hui de ces ouvertures à la concurrence : elles dégradent les services publics, démantèlent les monopoles publics pour en faire des monopoles privés, se traduisent par une baisse de qualité du service public, de la sécurité des infrastructures et, le plus souvent, par une augmentation des coûts pour les usagers. La question des personnels des transports publics est également centrale. Leur statut public n'est pas un archaïsme du passé, mais bien le corollaire de salariés tournés vers un objectif de service public, notamment de ces principes fondateurs : égalité, continuité, mutabilité et accessibilité. Aujourd'hui, vous proposez de dynamiter ce système en organisant le dumping social dans ce secteur, préconisant ainsi une harmonisation vers le bas des garanties salariales et la fin programmée du statut spécifique. Nous ne participerons pas à ce gâchis ! Nous pensons bien au contraire qu'il conviendrait de réfléchir, y compris pour aider et accompagner les collectivités dans leurs nouvelles compétences, à la création d'un opérateur public du transport urbain, à l'échelle nationale, qui permettrait de faire prévaloir les enjeux d'intérêt général sur ceux du privé privé et la complémentarité des modes plutôt que leur mise en concurrence. Dernier point : nous sommes absolument opposés à l'ajout en commission de l'allongement de la période de déclaration individuelle de grève.

Je me dois en effet de donner les raisons pour lesquelles nous devons rejeter cette motion tendant à opposer la question préalable, mais je dois, à la vérité, reconnaître que l'objet de cette motion est assez convaincant. Malheureusement, pour ses auteurs, convaincant ne veut pas dire convaincu ! Le résultat de ce paradoxe, c'est que je vais consacrer mon intervention à expliquer pourquoi les auteurs de la motion ont souvent raison, grief par grief, pour finalement vous demander, mes chers collègues, de ne pas la voter. Sur la forme, d'abord, les auteurs de cette motion nous rappellent avec malice toute l'étrangeté qu'il y a à débattre de ce projet de loi d'orientation des mobilités, alors même que nous sommes en plein grand débat national. Leur remarque est tout à fait justifiée : légiférer aujourd'hui, c'est, disons-le, faire peu de cas de ce grand débat national, faire peu de cas de la colère exprimée par les Français et c'est, enfin, faire peu de cas de l'aptitude des Français à donner leur avis sur une politique publique. Si le Gouvernement pense qu'il peut faire l'économie de la démocratie directe après avoir enjambé le Parlement- et le verbe « enjamber » est avantageux ... -, grand bien lui fasse ! Mais, dans ce cas, il eût été plus sage de ne pas convoquer nos compatriotes à cette grande procession républicaine. Toujours en ce qui concerne la concomitance entre le grand débat d'un côté et l'examen de ce projet de loi de l'autre, l'effet est d'autant plus maladroit que le détonateur des mouvements sociaux que nous avons traversés a été la hausse des prix des carburants. La crise des « gilets jaunes », bien qu'aujourd'hui envisagée comme une crise sociale ordinaire, est au départ une crise de la mobilité : mobilité sociale, certes, mais mobilité spatiale d'abord. Voilà pourquoi il me semble légèrement anachronique d'examiner ce projet de loi avant même l'issue du grand débat, ... Très bien ! ... mais soit ! Grief suivant exposé par les auteurs de la motion : le recours aux ordonnances. Difficile, là encore, de ne pas leur donner raison

En ce qui concerne le recours à un cabinet privé pour la rédaction de l'étude d'impact, le journal, dans un article du 29 novembre 2018, nous a indiqué que l'appel d'offres évoquait également l'exposé des motifs. Je ne crois pas que cette possibilité soit de nature à remettre en cause l'examen de ce texte ; en revanche, elle nécessite une clarification de la part du Gouvernement sur l'objet exact de l'appel d'offres. À titre personnel, je ne crois pas que nous assistions ici à un cas flagrant de méconnaissance de l'article 39 de la Constitution ni à une entorse aux dispositions organiques de la loi du 15 avril 2009. Reste que cela vient s'ajouter à une phase d'élaboration du projet de loi pour le moins laborieuse. Si ce processus d'élaboration a débuté dès la mise en place des Assises nationales de la mobilité, qui se sont tenues du 19 septembre au 13 décembre 2017, la phase de rédaction s'est, pour l'essentiel, achevée en août dernier avec la transmission d'une première version de l'avant-projet de loi au Conseil d'État. Une saisine rectificative a été adressée en octobre. Dans les deux cas, nous n'avons pas eu connaissance de son avis. L'avis du 15 novembre nous sera finalement transmis avec retard. Entre-temps, nous avons pu disposer des avis pour le moins réservés du Conseil national d'évaluation des normes et du Conseil économique, social et environnemental. Mais le Gouvernement décida, après que ces avis eurent été rendus publics, de modifier son projet de loi avant son passage en conseil des ministres pour s'adapter- je crois qu'il n'y a pas d'autre raison -au mouvement des « gilets jaunes Ont ainsi été retirées du projet de loi la création des péages urbains, qui devaient voir le jour dans les communes de plus de 100 000 habitants, la suppression de l'obligation d'une part minimale de véhicules à faibles émissions pour les entreprises et, enfin, la consécration législative du Conseil d'orientation des infrastructures. Voilà pour les principales, car la liste est bien sûr très incomplète. La phase d'élaboration du projet de loi ne s'est pas arrêtée là, puisque, dans une lettre rectificative du 20 février, le Gouvernement a souhaité procéder à l'ajout de six nouveaux articles. Heureusement pour vous, madame la ministre, notre rapporteur est un homme plein de bienveillance. Les auteurs de la motion ont d'ailleurs eu l'élégance de saluer son travail, qui, comme je viens de le préciser, n'a pas été rendu facile. Dans l'objet de la motion, il est notamment question de son travail sur le financement des infrastructures de transport. C'est justement le point que je veux aborder à présent.

Nos collègues évoquent la sanctuarisation des ressources de l'Afitf proposée par le rapporteur. J'ajouterai à cela l'affectation intégrale de la hausse de TICPE prévue par la loi de finances pour 2015 au financement des infrastructures de transport. Toujours en matière de financement des infrastructures, et toujours en ce qui concerne les faiblesses bien réelles de ce projet de loi sur ce point, nos collègues du groupe CRCE estiment que la question des investissements « reste reste posée afin de permettre un niveau d'investissement à la hauteur des besoins et pour le moins au niveau du scénario 3 présenté par le comité d'orientation des infrastructures Sans le savoir peut-être, les auteurs de la motion nous donnent la meilleure raison qui soit de commencer l'examen de ce texte. À ce propos, je crois savoir que nombre de mes collègues, et ce quel que soit leur groupe politique d'appartenance, se réjouissent à l'avance de pouvoir trouver des solutions de financement innovantes.

Autre grief dans la motion : les enjeux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique sont insuffisamment pris en compte, puisque l'alternative promue face à la voiture individuelle reste l'usage de la route au travers de la notion de mobilité partagée, qui est placée au même niveau d'exigence que la mobilité propre. Comment s'opposer à cette réflexion ? J'ajoute, en ce qui me concerne, que si le texte évoque la mobilité partagée et la mobilité propre, il eût été loisible, toujours pour dépasser notre horizon, de s'intéresser à la non-mobilité. On y pense trop peu souvent, mais la clé de mobilité actuelle qui conditionne nos besoins en mobilité propre ou en mobilité partagée, c'est l'accroissement constant des besoins de mobilité. Nous sommes à l'âge du « zapping » territorial, c'est-à-dire que nos concitoyens travaillent dans un lieu A, consomment dans un lieu B et font leurs démarches administratives dans un lieu C. La solution n'est pas toujours de savoir comment se déplacer, mais peut-être pourquoi se déplacer. Pourquoi alors prendre la peine d'équiper notre pays en fibre optique ? À quoi bon le développement de la 5G si, en définitive, nous ajoutons à ces nouveaux flux électroniques les flux physiques de l'ancien monde ? Dernier point de la motion dont je voudrais vous parler : la dénonciation de la libéralisation des transports urbains en Île-de-France. Par principe, je n'y suis pas opposé, comme la plupart de mes collègues du groupe Les Républicains. Comme la plupart d'entre eux également, je souscris aux garde-fous qui sont aujourd'hui envisagés, quoique insuffisants pour nos collègues du groupe CRCE. Mes chers collègues, je l'ai confessé dans mon propos liminaire, je suis trop souvent d'accord avec mes collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Rejoignez-nous ! On nous demande d'examiner cette loi en plein grand débat national, qui devait servir de fondement aux prochaines politiques publiques. Cette loi qui a trop souvent recours aux ordonnances, ... Ce n'est pas normal ! ... cette loi dont les contours ont changé à deux reprises, cette loi que le Conseil d'État, le Conseil national d'évaluation des normes et le CESE n'ont pas jugée aboutie, cette loi, enfin, qui n'est pas financée. Malgré tous ces griefs et la pertinence de chacun d'entre eux, le groupe Les Républicains votera contre cette motion. Nous pensons qu'il faut poursuivre la délibération. Nous pensons surtout que, dans le contexte politique actuel, il ne serait pas opportun de laisser l'exécutif poursuive son dialogue avec une opinion déboussolée. Quel

Je n'ose imaginer que vous refusiez ce débat. Au reste, vous avez déposé 105 amendements ... Eh oui, ce texte porte une ambition forte pour la transition écologique, et nous pourrons débattre des différents leviers proposés Eh oui, ce texte porte une ambition forte pour le transport ferroviaire ! Voici quelques chiffres : 80 % des investissements de l'État et de ses opérateurs, dans la décennie qui vient, vont être consacrés au ferroviaire, tandis que la route représente 85 % des déplacements dans notre pays. Oui, ce texte crée un droit à la mobilité dans une logique de services adaptés aux besoins et afin de ne plus laisser sans solution ceux qui ne bénéficient pas d'un service ferroviaire ! Oui, ce texte crée un cadre social protecteur pour les agents de la RATP,

Les raisons de cette position sont claires : tout d'abord, parce que le processus d'élaboration de ce texte a débuté dès la mise en place des Assises nationales de la mobilité, qui se sont tenues à la ensuite, parce que concevoir les mobilités de demain pour réduire les fractures territoriales et sociales est un enjeu essentiel et urgent ; enfin, parce que prévoir des ressources crédibles, pérennes et transparentes était absolument nécessaire.

En effet, sur son initiative, la commission a inscrit le principe d'une sanctuarisation des ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dont le budget ne peut dépendre de recettes instables et fluctuantes comme celles des amendes radars. La commission a également fixé dans la loi le principe de l'affectation intégrale de la hausse de la TICPE au financement des infrastructures de transport. Elle a par ailleurs fait de la réduction des inégalités territoriales son objectif prioritaire. Nous sommes bien évidemment ici, au Sénat, très sensibles à cette démarche. Attribuer une partie du produit de la TICPE au financement des services de mobilité dans les territoires dont les ressources sont insuffisantes permettra la mise en place de vraies alternatives à la voiture individuelle et de rompre le cercle vicieux de la « double peine » des habitants de ces territoires, dont les revendications sont, ne l'oublions pas, à l'origine de la crise des « gilets jaunes ». C'est donc en C'est donc en examinant ce texte que nous pourrons garantir la soutenabilité financière des investissements de l'État dans les infrastructures de transport pour les dix prochaines années.

Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est le fruit d'un long travail, puisqu'il a été élaboré à la suite des Assises nationales de la mobilité, lancées il y a déjà un an. La question des mobilités sur l'ensemble de notre territoire est essentielle et déterminante pour la cohésion sociale, comme le montre le fait que le mouvement des « gilets jaunes » a été déclenché par une hausse de la fiscalité sur le gazole. Elle doit donc retenir notre plus grande attention. Ce texte n'est pas encore satisfaisant : nous pensons qu'il ne va pas assez loin sur certains points et nous regrettons qu'il ait été fortement réduit par rapport à ce qu'il était initialement. Nous regrettons notamment, comme cela a déjà été souligné, qu'il ne règle pas la question des financements.

permettant ainsi des évolutions remarquables du texte lors de son examen en commission. Le débat en séance nous offre une occasion d'en voter d'autres. Si le groupe socialiste est encore réservé sur ce texte, il est convaincu que le débat doit avoir lieu. Après un long travail approfondi, des avancées obtenues en commission et d'autres peut-être à venir, il serait regrettable de le différer. Adopter cette motion reviendrait à renoncer à convaincre et peut-être à réduire notre propre parole. Or nous avons des propositions constructives à faire, sur lesquelles nous espérons être entendus. Nous souhaitons que ce débat puisse se tenir dans un esprit apaisé, sans céder à la provocation politique, comme la remise en cause des droits acquis, ce qui pourrait permettre, dans un esprit de conciliation, d'aboutir à des positions de consensus comme nous y sommes déjà parvenus en commission. Nous serons donc particulièrement vigilants sur tout recul du droit des salariés. Le groupe socialiste votera contre cette motion. Si nous comprenons, à certains égards, les arguments qui ont été développés à la fois sur le fond et la forme par nos collègues du groupe communiste, il nous semble nécessaire de débattre,

la première mobilité, c'est le spermatozoïde ; la dernière mobilité, c'est la dispersion des cendres. Entre les deux, c'est la vie ! Parlons de la vie

En parlant aujourd'hui de mobilités, nous montrons que notre approche a changé. Nous parlons même, cela reviendra dans le débat, de « droit à la mobilité », et je voudrais tout d'abord m'arrêter sur ce terme. Depuis 1982, nous avons beaucoup investi : en TGV, en autoroutes, en aéroports ... Nous avons changé la France et ses dynamiques de développement, grâce en particulier au TGV, les métropoles se sont affirmées, nous sommes sortis de la logique du, le célèbre livre de Jean-François Gravier paru en 1947. Mais, et il faut s'arrêter sur ce paradoxe, ce rééquilibrage permis par les infrastructures n'est pas ainsi perçu par tous nos concitoyens. Assèchement économique des territoires non métropolitains, étalement urbain et congestion des entrées de ville au petit matin, coût de la mobilité thermique disent une France en difficulté de mobilité, et la crise des « gilets jaunes » est dans toutes les têtes. Cette France à deux ou trois vitesses nous interpelle. Aussi, il est essentiel de souligner en introduction que, sans une politique de meilleure répartition des emplois, d'aménagement économique volontariste du territoire, les politiques de mobilité resteront en partie inefficientes, tentant de résoudre des problèmes dont elles ne sont pas à l'origine. Vous connaissez la vigilance et l'engagement du groupe du RDSE en faveur de cette exigence d'aménagement du territoire. En ce sens, nous regrettons que ce texte ne nous permette pas de discuter de tous les aspects de mobilité ayant un rôle clé d'aménagement du territoire, comme la gouvernance portuaire ou les aéroports de proximité, dont le rôle est précieux pour maintenir des entreprises dans des secteurs par ailleurs mal desservis- vous aurez noté que je peux même défendre des aéroports Cela étant dit, nous saluons, madame la ministre, le changement de discours que vous impulsez, cette priorité donnée aux mobilités du quotidien. C'est ainsi l'ouverture d'un nouveau cycle stratégique, qui doit participer de la cohésion nationale et, par ces financements, à la redistribution des richesses. le financement, justement, le texte n'est pas sans lacunes, et nous savons tous les centaines de millions d'euros qui manquent au budget de l'Afitf. Nous avons déjà, en commission, sur proposition de notre rapporteur, tenté de sécuriser une partie de ces financements en les dégageant de recettes aléatoires,

Plus largement, si nous soutenons évidemment la décentralisation des approches stratégiques, cela ne peut se faire sans un maintien d'une forte péréquation, d'une solidarité nationale forte, qui mériterait d'être mieux explicitée. Ce texte veut donner aux territoires plus de responsabilités au travers de la généralisation du rôle d'autorité organisatrice des mobilités. Nous ne pouvons que souscrire à cette approche décentralisatrice, au renforcement du couple région-intercommunalité. m'en féliciter, et le parallèle est évident avec la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, votée sous le précédent quinquennat, qui avait aussi renforcé ce même couple pour l'action climatique. En tant que président du groupe de travail « gouvernance » du débat national sur la transition énergétique, nous avions justement porté cette même proposition du tandem région-intercommunalité. De ce fait, le rapprochement entre les plans Climat les plans de mobilité est assez évident, et je remercie le rapporteur Didier Mandelli d'avoir accepté les amendements tendant à renforcer cette articulation. Je crois d'ailleurs que nous sommes nombreux, sur ces travées, à le remercier, lui qui a fait preuve d'une grande ouverture pour intégrer au texte des amendements venant de tous les groupes. À propos de l'action contre le dérèglement climatique, ce texte reste encore très timide sur plusieurs points clés : les moyens de ramener le transport de fret vers le rail et la perspective d'interdiction de vente à l'horizon de 2040 des véhicules thermiques neufs. Sur ce dernier point, le recul de l'État par rapport au plan Climat, puisque cet horizon est cité non plus dans la loi, mais simplement dans son préambule, ne peut que nous inquiéter. Cela ne donne pas aux constructeurs automobiles une perspective claire pour s'engager résolument dans cette mutation, ce qui détonne par rapport aux autres pays européens. fin de la commercialisation des véhicules thermiques est prévue pour 2030 au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande- et même en Inde -et pour 2040 au Royaume-Uni et en Espagne. Notre industrie automobile doit être engagée résolument dans cette mutation pour ne pas être marginalisée demain. Elle a donc besoin de signaux très clairs de la part de l'État. Cette réduction hautement nécessaire de nos émissions de gaz à effet de serre passe aussi par les nouvelles mobilités, même si elles ne répondent pas à tout : un bouchon de véhicules autonomes reste un bouchon, avec des véhicules à l'arrêt Aussi, nous devons rester volontaristes dans les signaux donnés aux modes de transport doux, notamment le vélo, en étant néanmoins conscients que leur développement et leur présence massive dans l'espace public appellent de nouvelles régulations. Le Sénat a fait oeuvre utile en développant quelques facilités pour les cyclistes dans les trains ou les parkings ; il serait dommage, madame la ministre, que le Gouvernement revienne en arrière sur certaines de ces modestes avancées. Nous serons donc vigilants. Les deux semaines qui s'ouvrent doivent nous permettre d'améliorer encore ce texte, qui nous semble néanmoins aller dans le bon sens. Le groupe du RDSE devrait donc très largement le soutenir. La parole

Ces collectivités sont les plus à même de prendre des dispositions permettant d'établir une mobilité vraiment durable et crédible. C'est donc une très bonne idée de décentraliser davantage ; les territoires de ce pays peuvent faire beaucoup, mais pas sans moyens. Ces derniers sont à la fois juridiques-

Nous nous félicitons, à cet égard, de la place qui a été accordée au vélo. La France devait se doter des moyens nécessaires au développement de l'usage de la bicyclette. Nous avons beaucoup de retard sur nos proches voisins européens ; je penche aux Belges, aux Hollandais aux Allemands. Les Français seront davantage incités à devenir cyclistes : la création de stationnements sécurisés pour vélos et de parcours cyclables d'envergure au travers du schéma national des véloroutes sera un élément décisif.

De nombreux points complémentaires pourraient être relevés. Je pense, par exemple, à la place de l'hydrogène dans la mobilité. Il n'y a pas de raison pour que le train à hydrogène ne circule pas encore sur nos lignes, alors qu'il est déjà en service en Allemagne. L'hydrogène est une énergie qui a de l'avenir ; j'en suis profondément convaincu. Je pense, évidemment- madame la ministre, vous ne m'en voudrez pas -, à l'avenir du canal Seine-Nord-Europe. Est-il vraiment nécessaire de changer, par la loi, le statut de l'établissement public ? J'ai vu que le Conseil d'État en doutait.

Nous croyons beaucoup à l'intermodalité dans le domaine de la mobilité, notamment collective. La diversité des réalités de notre pays appelle une pluralité de solutions. La parole

à en croire certains esprits bornés- c'est le qualificatif qui leur convient -, l'humanité serait renfermée dans un cercle de Popilius qu'elle ne saurait franchir, et condamnée à végéter sur ce globe sans jamais pouvoir s'élancer dans les espaces planétaires Il n'en est rien ! On va aller à la lune, on ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York, facilement, rapidement, sûrement, et l'océan atmosphérique sera bientôt traversé comme les océans de la lune ! » Voilà ce qu'écrivait Jules Verne au XIX siècle. En 2019, dans notre pays, nous nous interrogeons encore, certes, sur la réalité des voyages planétaires, mais bien davantage sur les trajets, les déplacements et les mobilités du quotidien. Cette question, je l'évoquais il y a encore quelques jours à Anor. Outre que cette charmante commune de l'Avesnois a la particularité d'être le point culminant du département du Nord, ses 3 300 habitants rencontrent aujourd'hui bien des difficultés dans leurs mobilités du quotidien, qu'il s'agisse de l'emploi, de la santé, des loisirs ou encore de la vie familiale. Anor n'est, hélas ! pas un cas isolé dans notre pays et témoigne bien des difficultés auxquelles se heurtent nos concitoyens, par trop souvent « assignés à résidence ». « Mobilité, mobilités », nous disent depuis plusieurs semaines nos concitoyens ; il n'est pas une seule rencontre qui se soit tenue dans le cadre du grand débat national dans laquelle ce thème ait été abordé, que l'on soit en ville ou à la campagne. En effet, le besoin de mobilité est réel le besoin de mobilité partagée, de mobilité fiscalement et socialement juste, mais aussi et surtout le besoin d'une mobilité pensée à l'aune des enjeux climatiques. Nos concitoyens veulent pouvoir vivre la mobilité, mais une mobilité qui soit pensée, organisée, accessible, pratique et aussi de plus en plus propre. projet de loi d'orientation des mobilités prend sens dans la France de 2019 ! Nous commençons l'examen d'un texte qui- nous l'espérons tous, quelles que soient nos convictions respectives -doit faire date et ouvrir des perspectives positives pour nos concitoyens. Le Sénat a oeuvré dans ce sens. Qu'il me soit permis de féliciter notre rapporteur, Didier Mandelli, pour la qualité du travail mené dans un souci permanent d'associer tous les commissaires à ce texte.

On doit évidemment évoquer les nouvelles infrastructures, mais aussi et surtout l'entretien et la remise à niveau du patrimoine existant, alpha et oméga de toute mobilité réussie, qu'elle soit pédestre, cyclable ou automobile. Ne nous trompons pas de combat en pointant du doigt l'automobile, cette bagnole devenue le mal du siècle, mais appelée demain à un nouvel avenir dans le cadre de ce que nous sommes nombreux ici à appeler de nos voeux : la fin du moteur thermique et le recours aux énergies décarbonées. La question des infrastructures est essentielle, tout comme la question de la gouvernance et l'assurance qu'il n'y ait plus, demain, de « zones blanches » de mobilités. Permettre aux collectivités territoriales de se saisir pleinement de la compétence mobilité, c'est la garantie pour nos concitoyens de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, et là est l'essentiel. Encore faut-il, pour ce faire, que les collectivités en aient les moyens et que ces chantiers soient menés dans des délais que nous qualifierons de raisonnables, au regard des renouvellements qui interviendront notamment en 2020. En matière de mobilités, il nous faut aller vers l'idéal et comprendre le réel ; je sais, madame la ministre, que ce point de vue Nous aurons l'occasion d'évoquer ce sujet à l'occasion de nos débats, mais nous partageons tous ici la même envie : donner aux collectivités les moyens de réussir la révolution, les révolutions des mobilités. N'ayons pas peur des mots : nous parlons d'une véritable révolution des usages et de révolution climatique en tentant de lutter efficacement contre la pollution de l'air. Avec la loi d'orientation des mobilités, nous disposerons demain d'une boîte à outils qui doit permettre, avant toute modélisation, d'expérimenter des modes de transport dont on a parfois tendance à penser, à tort, qu'ils ne sont pas faits pour nous, qu'ils ne sont pas adaptés aux contraintes du monde moderne.

contrairement à des idées trop souvent reçues, le vélo du quotidien n'est pas réservé aux habitants de plats pays ou aux citadins. La pratique du vélo, et notamment du vélo à assistance électrique, doit être encouragée au travers de diverses mesures. Je pense non seulement

Le Sénat est au coeur des mobilités et des mobilités douces : nous devons en faire la démonstration. Garantir le droit à la mobilité du quotidien, c'est permettre à toutes et à tous de se déplacer librement, sans contrainte aucune, en encourageant toutes les formes de mobilité et en incitant nos concitoyens à tendre vers une mobilité partagée.

Le sujet des mobilités est décidément passionnant, car, en définitive, il structure notre société. Avec ce texte, il peut préfigurer ce nouveau contrat social auquel bon nombre de nos concitoyens aspirent et dont la nécessité est plus qu'avérée dans un monde en permanente évolution. Notre responsabilité est immense, pour aujourd'hui, mais aussi et surtout pour demain et après-demain, dans tout le champ des mobilités, sans oublier- cela a été dit -le ferroviaire ou encore le secteur fluvial, que nous ne voulons plus voir comme un chef-d'oeuvre en péril. Notre responsabilité est immense, et le Sénat doit être au rendez-vous. Il l'est d'ailleurs, à en juger par le nombre d'amendements déposés sur ce texte, témoignant d'une appétence féroce pour le sujet.

Est maintenant venu le temps de l'action et des solutions. Ces dernières s'inscrivent dans le cadre d'une volonté dont nous ne doutons pas. Bien sûr, il reste encore quelques forteresses à prendre, mais c'est ensemble que nous y parviendrons. Nous ne pouvons plus attendre, car nos concitoyens ne comprendraient ni ne pardonneraient. Nous ne pouvons plus attendre, car l'urgence climatique est là, et l'affirmation, dans la loi, de la fin de la vente des véhicules thermiques pour 2040 est un marqueur fort qu'il nous faut confirmer. L'urgence climatique, nous devons y répondre avec ce texte de loi, et les outils ne manquent pas : les zones à faibles émissions, les énergies propres, le déploiement du vélo sont autant de points saillants sur lesquels nous ne pouvons pas transiger et qui appellent une prise de conscience collective ; autant d'enjeux que nous examinerons dans les prochains jours et qui rendent ce texte indispensable.

Merci

Nous aurions préféré l'examiner au printemps dernier, en même temps que la réforme ferroviaire : ce choix aurait été plus cohérent. Nous aurions préféré l'examiner dans sa version initiale, à 220 articles, avant que les réunions interministérielles ne le vident de sa substance et particulièrement de ses financements Entre-temps, le mouvement des « gilets jaunes » est venu rappeler l'enjeu primordial que constitue la mobilité pour nos concitoyens. Dans notre pays, l'urbanisme a été façonné par la voiture, qui relie de plus en plus des zones-dortoirs délaissées et des métropoles encombrées.

votre politique n'est que la continuité de ce mouvement, à une exception près : la prise en compte du fait qu'il est indispensable de sortir de l'ère du « tout-voiture individuelle ». Oui, mais comment ? Votre projet de loi ne répond que très partiellement à la question. La raison en est simple, et Gorz nous la donnait dès 1973 l'alternative à la bagnole ne peut être que globale. Car pour que les gens puissent renoncer à leur bagnole, il ne suffit point de leur offrir des moyens de transports collectifs plus commodes : il faut qu'ils puissent ne pas se faire transporter du tout parce qu'ils se sentiront chez eux dans leur quartier, leur commune, leur ville à l'échelle humaine, et qu'ils prendront plaisir à aller à pied de leur travail à leur domicile- à pied ou, à la rigueur, à bicyclette. » Nous en sommes très loin. Je ne reprendrai pas l'excellente démonstration de ma collègue Éliane Assassi pour rappeler que presque rien dans ce texte ne concerne les transports collectifs- demeurent pourtant la colonne vertébrale des mobilités -, si ce n'est l'ouverture à la concurrence de la RATP, qui fragilisera un peu plus nos capacités à entretenir et développer le réseau ferré francilien. Rien pour le rail- la question des lignes régionales est renvoyée à un énième rapport ! Rien pour le fluvial, ou presque ! Ce texte renonce d'emblée à l'ambition qui devrait être la sienne : restructurer notre réseau de transport, alors que pèse sur nous l'épée de Damoclès du changement climatique. d'une boîte à outils dans laquelle manqueraient les outils essentiels. Ce projet de loi n'est pas dénué d'intérêt pour autant, particulièrement dans la version que nous propose la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, qui l'a sérieusement musclé. Je salue à ce titre le travail de notre rapporteur, Didier Mandelli, qui n'a pas ménagé son effort et qui a pris soin d'associer l'ensemble des forces politiques à la rédaction de ce texte. Le projet de loi contient ainsi quelques dispositions intéressantes pour développer la pratique du vélo et des mobilités actives. Elles méritent toutefois d'être complétées, et plusieurs groupes le proposeront durant les débats. Aucun maire ne se plaindra de pouvoir réguler et mettre à contribution les entreprises de, qui inondent les trottoirs de vélos et de trottinettes électriques. Sur ce point également, il convient de conserver la rédaction du Sénat. S'ils ne sauraient remplacer les transports en commun en zone urbaine, le covoiturage et l'autopartage peuvent, en zone rurale, représenter des solutions de déplacement intéressantes pour limiter l'usage de la voiture personnelle. Ils sont également le seul débouché viable de la voiture électrique, qui ne peut qu'être partagée pour remplir son ambition écologique. Là aussi, nous invitons le Gouvernement à aller plus loin à l'occasion du débat parlementaire. pour lutter efficacement contre la pollution, dont on vient d'apprendre qu'elle tue en fait plus que le tabac- elle cause 67 000 décès par an dans notre pays -, il faut, sans mauvais jeu de mots, passer la seconde. Pour être efficace, le dispositif des zones à faibles émissions doit être renforcé et élargi à toutes les communes de plus de 50 000 habitants. Il faut également réintroduire dans le texte la fin des véhicules thermiques d'ici à 2040. Il faut aider les communes à développer leurs axes cyclables et des solutions non polluantes pour les livraisons dans le dernier kilomètre. Cet effort passe également par le nouveau « forfait mobilités », dont nous saluons la création, mais qui, pour atteindre son but, doit être cumulable avec un abonnement de transports en commun et rendu obligatoire, afin que chaque salarié puisse en bénéficier. Voilà un moyen efficace pour développer l'intermodalité que nous appelons tous de nos voeux Voilà un moyen efficace pour diminuer quelque peu le coût de la mobilité et apporter un début de réponse aux revendications des « gilets jaunes » ! Mes chers collègues, sans doute aurait-il fallu, pour ce faire, attendre les conclusions du grand débat. Nous avons tenté de les anticiper en vous proposant non seulement cette solution, mais également une prise en charge accrue des abonnements de transports en commun pour les salariés au SMIC. Nous vous proposerons aussi de renforcer la démocratie dans la gouvernance des AOM, en y associant les syndicats de personnels et les associations d'usagers : ce que nous rappelle le mouvement social en cours, c'est que, pour gouverner, il faut partir des besoins de la population dans tous les territoires. Les gouvernements successifs ont eu tendance à l'oublier de nos amendements ne comblera pas toutes les lacunes de ce texte, mais elle permettra de lui donner une densité supplémentaire et d'apporter davantage de réponses aux défis de la mobilité du XXI siècle. C'est le minimum que nos concitoyens sont en droit d'exiger de la première grande loi relative aux transports depuis près de quarante

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est peu de dire que, depuis 1982 et la promulgation de la LOTI, une nouvelle donne pour les mobilités et le transport dans notre pays se faisait attendre. Élu du monde rural, je constate chaque semaine dans mon département de la Dordogne les difficultés de nos concitoyens à se déplacer. Pour ceux qui n'ont d'autre solution que d'utiliser leur voiture au quotidien, les choix politiques sont sensibles : la colère déclenchée par la hausse de la fiscalité sur le gazole et relayée par les « gilets jaunes » exprime un sentiment d'abandon très prégnant dans ces « zones blanches » de la mobilité. Dès lors, ce projet de loi vise un objectif louable : renforcer les moyens pour les mobilités du quotidien et dégager des marges de manoeuvre pour les collectivités afin de s'en emparer.

Dès lors- c'est un peu son péché originel -, le texte étudié en commission présentait plusieurs lacunes importantes, en particulier s'agissant des financements pérennes dédiés aux infrastructures. Vous avez vous-même concédé le besoin de trouver 500 millions d'euros supplémentaires à partir de 2020 pour garantir les ressources de l'Afitf. sujet, je tiens à saluer l'important travail du rapporteur Didier Mandelli, ... Très bien ! ... qui a su proposer un grand nombre de dispositifs de compromis pour compenser les carences identifiées.

j'approuve la philosophie du texte, consistant à faire des régions les chefs de file des mobilités dans notre pays, aux côtés des EPCI. Mais ces derniers doivent pouvoir bénéficier de marges de manoeuvre plus grandes pour se saisir, eux aussi, des compétences dédiées. La mise en oeuvre d'un versement mobilité plus souple et plus strictement conditionné à l'organisation de services réguliers répond à cet impératif, de même que l'affirmation des contrats de mobilité comme outils adaptés pour inciter plus encore au conventionnement. Je me félicite tout particulièrement de l'attribution d'une partie de la TICPE aux mobilités dans les territoires peu denses. Cette solution permettra aux AOM de compléter le produit d'un versement mobilité insuffisant dans certains départements, comme le mien,

Ce type de mesure rejoint notre volonté de vous proposer plusieurs nouvelles pistes de financements innovants, tant au profit de l'Afitf que des collectivités territoriales, afin de mieux répondre au défi des mobilités de demain. Avec mes collègues du groupe socialiste, nous défendrons plus d'une centaine d'amendements, qui tendent à aller encore plus loin au profit des collectivités et des initiatives locales mobilité additionnel et transitoire pour financer localement des projets d'infrastructures ; fléchage d'une partie de la TICPE vers les EPCI développant des services de mobilité sobre et faiblement émettrice ; ou encore meilleure association des départements, détenteurs de la compétence de gestion des routes, aux politiques de mobilité. Certes, notre proposition d'instaurer une redevance kilométrique pour les poids lourds, assortie d'une suppression de la taxe à l'essieu, n'a pas passé le couperet de l'article 40, mais elle reflète notre volonté de doter le pays d'un dispositif conforme aux règles européennes visant à faire contribuer les transporteurs étrangers au financement de notre réseau routier national, sans les discriminer sur la base d'arguments nationalistes contestables. Nous serons très attentifs au débat que suscitera notre proposition de grand emprunt national au profit des infrastructures de transport. En effet, nous avons l'audace de penser, dans la lignée de plusieurs économistes de renom, que le financement des mobilités durables, comme celui de la transition énergétique, doit bénéficier d'un véritable plan d'investissement sur le long terme.

de loi d'orientation des mobilités, tant attendu par les acteurs du secteur et les citoyens, est à l'étude. Qui plus est, la première lecture commence devant le Sénat. Le fait est suffisamment rare pour être souligné pour la confiance que vous témoignez à la Haute Assemblée, pour votre qualité d'écoute lors des différents échanges et pour les nombreuses phases de concertation menées en préparation de ce projet de loi, je tiens à vous remercier tout particulièrement. Je remercie

également remercier les organismes professionnels, associations d'élus ou de citoyens, les entreprises, les collectivités avec qui nous avons eu des échanges constructifs durant nos travaux pour améliorer un texte qui se devra de faire référence durablement.

vous le savez, ce projet de loi est essentiel, car la mobilité est absolument indispensable à tous les actes de la vie. Elle concerne tous les citoyens, quels que soient leur statut, leur âge, leur lieu de résidence, qu'ils soient femme ou homme, actif ou retraité, demandeur d'emploi ou étudiant. Que l'on vive en ville ou à la campagne, dans une métropole ou une commune isolée, on a toujours besoin de se déplacer pour étudier, travailler, se soigner, faire des courses, se cultiver ou aller voir des amis. Même pour utiliser un espace de, il faut se déplacer.

Le maître mot, l'objectif principal, l'enjeu, c'est bien qu'il n'y ait plus aucune « zone blanche » de mobilité sur notre territoire. Voilà pourquoi nous devons engager une réflexion sur la notion d'équité, notion différente de l'égalité stricte, entre tous nos territoires et sur la nécessité de trouver des solutions adaptées à la réalité concrète du terrain. Plus que jamais, cette situation nous interroge quant aux solutions de mobilité pour tous, qui, de manière évidente, n'excluent pas la voiture, même si elle de moins en moins sacro-sainte ; quant aux solutions en fonction des territoires ; quant à l'impérieuse nécessité de créer un cadre propice au dialogue, à la décision et au financement entre les différentes strates administratives concernées. Ce projet de loi nous conduit également à nous interroger sur le partage des données. Cherchant constamment à me mettre en situation d'usage et empruntant régulièrement les transports publics, je considère que tous les travaux entrepris dans la logique du MaaS- -vont dans le bon sens s'agissant déjà d'intermodalités, des mobilités actives au, de la marche à pied aux navettes autonomes. Le transfert des données à l'autorité organisatrice est alors une condition de la pertinence de l'outil. Tandis que plane l'ombre de GAFA, il est de notre devoir de définir les conditions du succès de ces nouveaux services, en s'assurant qu'aucun prestataire privé ne puisse en tirer un avantage concurrentiel. L'intérêt général doit primer les intérêts particuliers. Malgré toutes ces bonnes intentions, nous déplorons qu'au fil des jours, ou des arbitrages interministériels, ce texte tant attendu se soit vidé petit à petit de sa substance au point de manquer singulièrement d'ambition, notamment au regard de l'enjeu climatique et du développement durable. loi a été dangereusement édulcoré pour ne pas faire de vagues dans le contexte politique actuel. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire de l'amender. Le grand nombre d'amendements

Il est également dommage d'examiner ce projet de loi en sachant que certaines de ses lacunes ne pourront être gommées à court terme ; parce que des sujets, pourtant essentiels, demeurent à l'étude au sein du ministère- je pense à la péréquation du versement mobilité ou encore à la taxe pour les poids lourds étrangers

La présentation récente du budget de l'Afitf n'est pas parvenue à nous rassurer. Je fais partie de ceux pour qui les ressources issues des mobilités, la TICPE notamment, doivent être fléchées vers les mobilités. Les taxes, péages, impôts et autres redevances ont alors un sens, une réalité objective facilitant leur acceptation. Imaginer un financement d'infrastructures prioritaires en les corrélant à la productivité des radars, sachant que l'Afitf est la dernière servie, relève plus du non-sens que de la stratégie. Pour conclure, alors que j'évoquais à l'instant les problèmes de financement, je voudrais vous lancer un défi, fonctionnement a amené les collectivités locales à revoir leur organisation, à remettre en question les process, à améliorer leur politique d'achats, dans un souci constant d'économie.

Madame la ministre, ils attendent du Gouvernement, et par la force des choses de nous, la mise en oeuvre d'une politique volontariste pour un meilleur aménagement du territoire. Cet objectif nous oblige. Malheureusement, le texte initial ne plaçait pas cette préoccupation au sommet des priorités du projet de loi et, comme ce fut le cas d'ailleurs avec la réforme

Ce projet de loi comporte cinq titres, mais l'un d'entre eux a fait l'objet d'une attention particulière de la part de notre commission : celui relatif à la programmation des investissements de l'État dans les infrastructures de transport. Cette programmation s'appuie essentiellement sur le rapport du comité d'orientation des infrastructures publié en février 2018, qui présentait trois scénarios en matière de priorités d'investissements. Madame la ministre, vous avez opté pour le scénario n° 2. Je ne Je ne souhaite pas m'attarder sur les difficultés de financement clairement identifiées et corrigées par notre commission, qui a prévu des ressources crédibles et pérennes pour financer cette réforme. Toutefois, je veux vous dire que le choix de ce scénario est, de mon point de vue, la plus importante marque de renonciation à l'ambition initiale du texte, à savoir « offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui », comme l'indique la première phrase de l'exposé des motifs.

: celui de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, la POCL. Né en 2007 et toujours inscrit dans le Grenelle de l'environnement, ce projet, comme d'autres, ne cesse de faire l'objet d'une procrastination étatique.

Nous sommes d'accord pour privilégier la rénovation et la modernisation des lignes existantes, à l'image de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, dite

est très attendu par nos territoires et nos concitoyens. Le travail de la commission a notamment permis de mettre en évidence certaines difficultés de financement. Il est évident que de nouvelles ressources vont devoir être trouvées.

que prévu par ce projet de loi, et celui qui a été publié le 27 février dernier par l'agence elle-même. La France a depuis longtemps besoin d'investissements importants pour maintenir et développer ses infrastructures de transport ; ce n'est pas une nouveauté. La situation actuelle de nos territoires n'est pas satisfaisante : beaucoup d'entre eux ont toujours besoin d'être désenclavés, d'où la pertinence de ce projet de loi.

On peut en effet compter sur leur ingéniosité pour imaginer des solutions pragmatiques, mais il faudra mobiliser des fonds suffisants pour que celles-ci Certains territoires ne nous ont d'ailleurs pas attendus. À ce titre, l'ouverture des données est une très bonne chose. Des solutions de mobilité existent parfois déjà, mais elles ne sont pas assez utilisées, faute d'être suffisamment connues du public. On peut aussi

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, s'il est difficile de prédire quelle sera la place de ce texte dans l'histoire des transports de notre pays, nul ne peut contester que, par son intitulé, il marque une rupture avec un monde organisé sous l'autorité de l'État. Vous me permettrez de concentrer mon propos sur le sujet de l'État stratège.

Lyon-Turin s'inscrit donc clairement dans l'enjeu méditerranéen de demain. Lancée par Cavour en 1857, avant que la Savoie ne devienne française, la construction de ce tunnel ferroviaire fut une première mondiale.

L'ambition politique française a été affichée très tôt, dès le traité de Turin de 2001, avec l'engagement du Président de la République de l'époque, Jacques Chirac, confirmé successivement par les présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande et, plus récemment, Emmanuel Macron. Vous-même, madame le ministre, avez rappelé que le tunnel transfrontalier et ses accès faisaient partie intégrante du traité transfrontalier relatif au Lyon-Turin ; je vous en remercie. L'actualité nous conduit à rappeler que le tunnel transfrontalier de 57,7 kilomètres, d'un coût de 8,6 milliards d'euros, est financé à 40 % par l'Europe, à 35 % par l'Italie et à 25 % par la France, alors que l'ouvrage est situé à 80 % sur notre territoire, au coeur des accès de la liaison Lyon-Turin, d'une longueur de 270 kilomètres. Avec ce tunnel de basse altitude, la France se mettra au niveau des infrastructures transfrontalières européennes de l'arc alpin, après les tunnels du Lötschberg, du Saint-Gothard et du Brenner.

de ces défis, j'ai deux questions précises à vous poser, madame le ministre. La première concerne les financements européens. Le Gouvernement italien a accepté la poursuite des travaux et des appels d'offres du tunnel transfrontalier, en saisissant Bruxelles pour renégocier les financements. en juin dernier, une proposition visant à renouveler le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE, en portant le cofinancement de l'Europe de 40 % à 50 % pour les projets liés aux liaisons transfrontalières. Le Lyon-Turin, qui relève de ces grands projets, est éligible à cette augmentation de taux pour le tunnel, mais également pour le financement des accès. À un moment aussi décisif pour ce projet, la France doit saisir cette occasion européenne.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, ce projet de loi part de constats inattaquables et répond à des objectifs auxquels on ne peut que souscrire le domaine des transports connaît une mutation profonde, les échanges se multiplient à grande vitesse, engendrant des dommages irrémédiables pour notre planète, qu'une grande partie de nos concitoyens voient s'allonger leurs trajets quotidiens, éprouvent un sentiment d'isolement, d'assignation à résidence, et ont besoin de moyens de déplacement plus efficaces et moins coûteux. En ce sens, nous saluons les mesures qui, dans ce texte, accompagnent la mue numérique, ainsi que les nouveaux usages, notamment le déploiement de modes de transport alternatifs, l'ouverture des données de mobilité dans le respect de la vie privée et le développement des services d'information sur les déplacements. Néanmoins, cette révolution ne doit pas être synonyme de régression sociale. Le Gouvernement a prévu la possibilité, pour les plateformes, d'établir une charte offrant de pseudo-droits aux travailleurs passant par leur intermédiaire sans être salariés. être salariés. Cette mesure est insuffisante, puisque facultative, et surtout elle instaure un dispositif au rabais, à l'entier bénéfice des plateformes, sans réelle protection des travailleurs. Il faut mettre fin à ce système ! C'est pourquoi nous voulons supprimer cette disposition et demandons la mise en place d'une branche professionnelle, ainsi que la garantie d'un salaire minimum. Le respect du droit du travail n'est pas une simple option, et, à cet égard, l'amendement qui vise à imposer un service normal garanti aux heures de pointe pendant les périodes de grève est à nos yeux inacceptable. Nous nous y opposerons fermement De la même manière, s'agissant de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus actuellement exploitées par la RATP, nous veillerons à la sauvegarde des conditions d'emploi des d'emploi des salariés et défendrons la mise en place d'un « sac à dos social », ainsi que la continuité des droits acquis, tout en prévoyant un haut niveau social La mobilité représente un enjeu fondamental en matière de cohésion et d'intégration sociales. Nous compléterons donc les mesures prévues pour accompagner davantage les personnes fragilisées et favoriser leur mobilité, ainsi que pour tenir compte du caractère insulaire des territoires ultramarins.

S'il comporte des mesures encourageantes, le texte présenté ne s'engage pas suffisamment dans la voie de la sortie du « tout-voiture ». Ainsi, le transport fluvial, écologiquement l'un des plus vertueux, est le parent pauvre de ce C'est là un énorme paradoxe : le trafic routier sature, engendrant nuisances et pollutions, alors que nos voies navigables, les plus longues d'Europe, sont largement sous-exploitées. En cela, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Trop timide, il donne le sentiment de prolonger une logique ancienne plutôt que de préparer le monde de demain, un monde décarboné dans lequel nos mobilités devront obligatoirement respecter notre environnement. Osons changer de paradigme ! Osons avoir de l'ambition Attelons-nous réellement à repenser l'organisation du travail pour limiter nos déplacements, avec des horaires décalés ou le télétravail, mettons fin à la vente de nouveaux véhicules thermiques, comme nous le proposons, et régulons le transport de marchandises autant de sujets essentiels sur lesquels ce texte fait l'impasse, tout comme sur ceux du transport aérien ou de l'avenir des petites lignes, pourtant cruciales pour la mobilité de nombreux citoyens.

Pour relever ce défi, nous proposerons à l'État de lever un grand emprunt : c'est plus que nécessaire pour accélérer la transition écologique.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, les Français sont plus que jamais en attente de solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie, faciliter leur mobilité, notamment en zones rurales. Eu égard à l'ensemble des recommandations émises par cette chambre et aux préconisations du Conseil d'orientation des infrastructures,

Mais quelle déception de devoir constater que cette mesure, inscrite à l'article 1, est le seul élément de la politique d'aménagement du territoire que nous attendions du Gouvernement ! Quelle déception nous avons éprouvée à la lecture d'un texte qui se focalise uniquement sur les mobilités électriques, et donc sur la voiture électrique Force est de constater que ce projet de loi ne répond pas aux attentes exprimées sur le terrain et qu'il ne va pas assez loin pour répondre aux défis technologiques, sociaux et environnementaux de l'avenir.

Pourquoi les petites lignes ferroviaires sont-elles absentes du texte, malgré leur importance capitale ? Pourquoi les collectivités territoriales ne bénéficient-elles pas de moyens pour assumer les nouvelles compétences que leur confère ce texte ?

était un jour comme les autres. À l'approche des fêtes de Noël, les familles se préparaient à se retrouver dans la chaleur de leur foyer. Mais ce jeudi 14 décembre 2017, à 16 h 03, les vingt-deux collégiens de Millas qui rentraient à la maison en car ont vu leurs vies basculer en une fraction de seconde. Leur bus s'est fait percuter de plein fouet par un TER en traversant le passage à niveau. Soudain, le chaos, l'obscurité ... Léana, onze ans, constate le drame : six de ses amis sont morts, quatorze autres blessés à jamais des images qui resteront gravées dans le corps et la mémoire de cette collégienne, ainsi que de toutes les personnes qui ont été touchées par ce terrible événement. J'étais présent, en cette nuit terrible, aux côtés des familles et des collégiens, face à ce bus coupé en deux, avec les élus, les représentants de l'État, les forces de l'ordre, les pompiers et les agents de la SNCF. Peut-on trouver les mots justes pour décrire l'effroi de toute une population devant la perte de six petits anges qui avaient toute une vie devant eux ? Lors du rassemblement en hommage à nos enfants décédés, vous étiez présente, madame la ministre, dix ans après le drame d'Allinges, en Haute-Savoie. Quel est le rôle d'un élu de la Nation ? Faire en sorte qu'un tel drame ne puisse jamais se reproduire ; réfléchir le plus efficacement possible à de dispositifs permettant de sécuriser les 13 000 passages à niveau français ; poser des actes. C'est pourquoi j'ai déposé, le 5 juin, une proposition de loi, dont j'ai souhaité qu'elle soit intégrée au texte élaboré par notre commission. J'espère de tout coeur que cette proposition de bon sens, composée de trois dispositifs, fera l'objet d'un vote unanime de la Haute Assemblée. Je remercie le président de la commission, M. Hervé Maurey, et le rapporteur, M. Didier Mandelli, de l'avoir accueillie favorablement. J'aurai l'occasion d'y revenir.

d'agir en adoptant ces dispositifs transpartisans. Madame la ministre, les élus que nous sommes, mon département et les familles endeuillées à jamais vous seront infiniment reconnaissants

Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 36 du règlement du Sénat, relatif à l'organisation de nos travaux. Je suis quelque peu surpris de l'usage extravagant fait de l'article 40 de la Constitution pour limiter l'exercice du droit d'amendement d'un parlementaire. Je suis surpris que mon amendement visant à dissoudre la société du Grand Paris au sein d'Île-de-France Mobilités ait été ainsi discrètement écarté. Comment la commission des finances peut-elle expliquer que la suppression d'un établissement public ayant coûté

doit assumer pleinement. Vous devez ainsi donner les moyens financiers nécessaires aux échelons locaux quand vous leur transférez des missions dans le cadre des expérimentations que vous souhaitez mettre en place. Par ailleurs, comme votre texte a pour ambition d'orienter les mobilités, il est essentiel qu'il marque la bonne direction. Cela consiste notamment à tenir compte des territoires et de leurs spécificités.

D'autres ont besoin qu'on tienne compte de leur réalité, qu'on ne leur impose pas des normes centralisées sans distinction, comme cela a été fait pour la limitation

Je conclurai en paraphrasant mon ami Rémy Pointereau : un pays qui n'investit plus est un pays qui se meurt

Partant de ce travail, vous avez cherché, madame la ministre, à construire une planification robuste et réaliste. Vos priorités méritent d'être soutenues. Je pense notamment aux noeuds ferroviaires saturés,

Vous l'avez souligné, madame la ministre, la question du financement est très liée au grand débat national qui s'achève. Le défi est de trouver des ressources en évitant d'augmenter la fiscalité, surtout pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture

comment aborder sereinement la question du financement des infrastructures et celle des objectifs des pouvoirs publics en la matière, alors même que la presse a annoncé, la semaine dernière, la suppression de 56 lignes et la fermeture de 120 gares ferroviaires ? Comment aborder sérieusement cette problématique, alors que la question des lignes de vie est renvoyée à un énième rapport qui sera rendu, bien entendu, après l'examen de ce projet de loi ? Le traitement de cette question devrait pourtant constituer l'un des engagements prioritaires de cette programmation : nos territoires ont besoin que soit conservé et renforcé le maillage ferroviaire de notre pays. Les déclarations d'intention qui sous-tendent cet article sont très directement démenties par la politique gouvernementale, ce qui entache la confiance dans les engagements pris. Par ailleurs, alors que répondre au défi climatique est présenté comme une urgence absolue et que des milliers de nos concitoyens se sont mobilisés samedi dernier, pourquoi renoncer à aborder la question du question du transport de marchandises, réduite par ce rapport à celles de la compétitivité des ports et des autoroutes ferroviaires ? Pourquoi faire des « mobilités partagées » l'équivalent des transports en commun, alors que le coût environnemental n'est évidemment pas le même ? Ce sont là autant de questions qui nous conduisent à nous interroger sur le modèle retenu par le Gouvernement. Après avoir promu le remplacement des trains par les « cars Macron »,

c'est tout l'esprit du projet de loi que nous examinons. Je souhaite appeler votre attention, madame la ministre, sur deux projets qui visent à atteindre cet objectif.

Cette desserte ferroviaire est indispensable pour gagner la bataille environnementale du ferroviaire contre l'aérien et le routier. Le GPSO est le maillon manquant de la grande vitesse européenne jusqu'à l'Espagne. C'est l'un des axes stratégiques du réseau européen pour relier la péninsule ibérique au reste de l'Europe par la façade Atlantique, tant pour le fret que pour le trafic voyageurs, d'autant que la ligne Dax-Espagne est envisagée comme une solution de transport écologique et durable, au regard des des 44 millions de tonnes de marchandises qui franchissent chaque année par la route la frontière entre la France et l'Espagne. En second lieu, madame la ministre, développer les mobilités du quotidien, c'est aussi l'esprit de l'étude sur l'amélioration de la desserte de Pau

Pourtant, toutes les collectivités concernées ont travaillé ensemble, voté des délibérations pour prévoir le financement de cette étude. Seul l'engagement de l'État reste à formaliser. Madame la ministre, nous avons déjà pu évoquer ce sujet ensemble. Je vous demande plus

Je regrette que nous ne puissions avoir ce débat, car il est essentiel pour nos mobilités, pour notre développement économique et pour l'aménagement de notre territoire. Depuis la réforme portuaire d'octobre 2008, le statut de grand port maritime s'est substitué à celui de port autonome. Ce statut regroupe néanmoins pêle-mêle des ports à vocation internationale au même titre que des ports placés sur des axes de trafic national. Or, concernant ces derniers, de nombreux élus locaux se prononcent depuis plusieurs années pour une plus grande implication des collectivités territoriales. Les grands ports maritimes restent, aujourd'hui, les derniers ports ayant pour obligation de conserver un statut d'établissement public placé sous la responsabilité de l'État, comme le permet l'article 22 de la loi NOTRe. Dans un rapport publié au mois de février 2017, la Cour des comptes rappelait l'urgence de trancher la question de la gestion des grands ports maritimes. Elle soulignait que la réforme des grands ports maritimes avait donné lieu à « une mise en oeuvre inégale, des effets modestes, une attractivité insuffisante ». À titre d'exemple, ce rapport mettait en évidence les difficultés financières du grand port maritime de Bordeaux, liées à un manque de vision stratégique territorialisée. Le transfert de la compétence portuaire à la région permettrait une meilleure association des partenaires économiques et industriels. L'État resterait néanmoins un acteur central pour l'accomplissement des missions régaliennes liées à la sécurité maritime et au contrôle des flux, ainsi qu'au titre de sa compétence en matière de dragage.

Ainsi, « le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales par des aménagements d'itinéraires existants » figure parmi les priorités retenues. Dans le département de la Loire, la mise à 2x2 voies de la route nationale 7 au niveau de Mably est indispensable pour désenclaver Roanne. Alors qu'il avait été prévu dans le contrat de plan État-région 2015-2020 de réaliser les études, les crédits nécessaires ne sont toujours pas débloqués. Cette opération n'apparaît pas clairement dans le rapport annexé. Madame la ministre, pouvez-vous me confirmer que les lignes génériques « Études amont » ou « CPER Route » permettront de répondre aux besoins ? ailleurs, vous proposez de rompre avec les « impasses d'une politique d'infrastructures tournée vers les grands projets et non financée depuis des décennies ». Je ne peux que saluer une telle orientation, qui, je l'espère, permettra de sortir d'une impasse dans laquelle nous nous trouvons depuis près de trente En effet, le projet de création d'une nouvelle autoroute, l'A 45, entre Saint-Étienne et Lyon a longtemps achoppé sur l'insuffisance du financement, si longtemps qu'il en est devenu obsolète et inacceptable au regard des impératifs de la transition écologique. C'est ainsi que vous avez annoncé, au mois d'octobre dernier, l'abandon du projet de l'A 45, ainsi que le préconisait le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron. Pour autant, la connexion entre les deux premières villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste largement problématique. Aussi je me félicite que l'exposé des motifs de ce projet de loi indique que « l'amélioration des déplacements entre Lyon et Saint-Étienne est une priorité » et que les 400 millions d'euros prévus initialement pour la réalisation de l'A 45 apparaissent dans le rapport annexé au titre du financement des projets alternatifs. Alors que le projet de l'A 45 a longtemps empêché toute réflexion collective sur ces liaisons, nous travaillons étroitement, avec mon collègue député de la Loire Régis Juanico et mes collègues du Rhône Gilbert-Luc Devinaz et Annie Guillemot, à une réponse conjointe à la concertation. Aujourd'hui, toutefois, certains élus des territoires concernés refusent de s'impliquer dans cette concertation, croyant que le projet de l'A 45 pourra être relancé. Afin qu'ils puissent avancer avec nous dans la construction d'alternatives, il conviendrait de formaliser l'abandon définitif de ce projet. Nous défendrons tout à l'heure un amendement en ce sens.

Féret, sur l'article. Madame la ministre, je souhaite évoquer la ligne nouvelle Paris-Normandie, la LNPN. Les objectifs de départ étaient ambitieux : augmenter la fréquence et le nombre des dessertes ferroviaires de la Normandie, réduire les temps de parcours et améliorer la qualité de service. Au-delà du transport de passagers et de marchandises, c'étaient bien l'aménagement de la vallée de la Seine, le développement économique par le désenclavement de la Normandie et la politique maritime de la France qui se jouaient. Force est de constater, à la lecture du volet relatif à la programmation de ce projet de loi, que tout cela n'est pas pour demain ... Même pour quelques sections jugées prioritaires, les opérations courraient au mieux jusqu'en 2037 ! De fait, pour les habitants de mon département,

égard à toutes les réserves émises sur la sincérité de la programmation financière développée dans le rapport annexé au présent projet de loi, je me dis que les usagers de la ligne Paris-Caen-Cherbourg, que je connais bien, ont encore bien des galères et des retards devant eux Madame la ministre, nous attendions un engagement fort de l'État, avec un échéancier ambitieux tenant compte des besoins de notre territoire et des usagers. Si l'Atlantique s'est rapproché de la capitale ces dernières années, la Manche reste de toute évidence une zone non prioritaire, totalement transparente.

cet après-midi ! Réduire les inégalités territoriales en renforçant l'accessibilité des zones rurales enclavées, améliorer la qualité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution et la congestion routière, accroître l'efficacité des transports de marchandises quatre objectifs pour cette programmation et cette stratégie en matière de mobilité auxquels je ne peux que souscrire. Je remercie le rapporteur de les avoir intégrés dès le début de ce texte ô combien important pour nos territoires en général, et pour l'Oise en particulier.

d'une infrastructure qui, à l'heure de la transition écologique, privilégie le transport ferroviaire, décongestionne l'A 1, donne accès aux Oisiens à un aéroport international et à une gare TGV, mais qui constitue surtout une porte d'entrée à la zone d'activité de Roissy-Charles-de-Gaulle, tout cela en six

que la robustesse et la capacité de la ligne TGV seront augmentées. Aujourd'hui, 40 TGV passent en pleine ville ; demain, il y en aura 120, 130 ou 140 ... C'est un sujet d'inquiétude pour les habitants.

Montpellier-Perpignan sont vraiment des projets structurants de développement du territoire, en particulier pour l'Occitanie. Je m'attarderai plus particulièrement sur le projet de ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, à propos duquel je suis intervenu ici même

sur l'Espagne et l'Europe n'a toujours pas été réalisée. J'ai été rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord franco-espagnol pour la réalisation de la ligne à grande vitesse transpyrénéenne Perpignan-Figueras.

que le Conseil de l'Union européenne vient de confirmer que « l'Europe veut s'assurer que son programme phare concernant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe continuera de financer les projets clés dans le domaine des transports, notamment ».

avancent au niveau national. J'ose donc espérer, madame la ministre, que vous donnerez un avis favorable à l'amendement n° 870, qui a été déposé par Angèle Préville et plusieurs sénateurs d'Occitanie.

unanimement apprécié. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, et particulièrement sur la section Rouen-Barentin. Ces projets figurent parmi les programmes d'investissements prioritaires.

pour une meilleure qualité de vie, et de renforcer l'efficacité et le report modal dans le transport de marchandises. La nouvelle gare de Rouen permettra d'améliorer les offres de déplacement du quotidien, d'accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, de contribuer à la cohésion des territoires et, enfin, de renforcer l'efficacité des transports de marchandises pour accroître la compétitivité des territoires et des ports.

très largement sous-dimensionnés au regard des besoins, qu'il s'agisse du réseau existant ou de l'infrastructure à créer. C'est la raison pour laquelle je tenais à intervenir cet après-midi

dans la continuité de l'intervention de mon collègue Jean-Pierre Vial lors de la discussion générale. L'État réaffirme, au travers de ce projet de loi d'orientation des mobilités, son engagement à réaliser le tunnel transfrontalier et il confirme l'intérêt stratégique de l'ouvrage sur les plans économique et écologique.

J'ajoute que, pour ce quinquennat, j'ai trouvé 10 milliards d'euros d'engagements non financés. Je suis tout à fait d'accord avec le sénateur Pointereau : un pays qui n'investit pas est un pays qui se meurt.

au renforcement des lignes ferroviaires autour des métropoles et au désenclavement, nous posons un acte fort en termes d'aménagement du territoire.

J'ajoute que la mise en service de la liaison Serqueux-Gisors permettra de sortir du trafic un certain nombre de trains de fret qui viennent perturber les circulations, et donc la régularité des dessertes, sur ces lignes normandes.

une infrastructure située en Île-de-France, sa modernisation est fortement attendue par toutes les régions qui bénéficient de TGV en interconnexion. Absolument ! Les travaux sur la section est démarrent cette année et se poursuivront, au titre du prochain contrat de plan, sur la section ouest. Évidemment, des protections phoniques seront mises

avec des dizaines de milliards d'euros promis dans tout le pays, à un exercice inédit et exigeant. Nous tenons nos engagements au titre de 2019 et nous aurons à débattre ensemble de la ressource que nous devrons dégager à partir de 2020. L'amendement

n'ont d'autre dessein que de recréer des monopoles privés autour des géants du BTP, au détriment des intérêts des usagers. En effet, partout où ce processus a été mis en oeuvre, les tarifs ont augmenté et le service rendu L'intérêt général est bafoué et les usagers sont considérés comme de simples réservoirs à dividendes pour les actionnaires de ces sociétés privées, puisqu'ils se trouvent dans une situation particulièrement captive. Les partenariats public-privé en matière d'infrastructures se sont également révélés particulièrement coûteux pour les deniers publics et, le plus souvent, le résultat est de piètre qualité. Nous considérons que ces politiques de vente du patrimoine historique de l'État, outil industriel majeur pour l'aménagement du territoire, tout comme le fait de confier les nouvelles infrastructures au privé, sont le signe de l'impuissance et du désengagement de l'État. C'est une politique de courte vue, dont l'unique vocation est de répondre aux injonctions de désendettement de l'État et

des zones les plus enclavées puissent bénéficier de conditions satisfaisantes d'accès aux services publics. C'est un élément déterminant, qui a joué un rôle moteur dans les mouvements sociaux de ces derniers mois.

que « les dispositions de portée générale, ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement, ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif ». Quel est l'avis de la commission est l'avis de la commission ? Il est vrai que les conditions climatiques ont un impact sur l'état de nos infrastructures, mais ce n'est pas le seul facteur : il y a aussi la densité du trafic, l'ancienneté du réseau, etc.

libellé : La parole est à M. Yves Bouloux. Cet amendement vise à compléter l'objectif d'amélioration des liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, en particulier les communautés urbaines.

En vue du respect de ses engagements climatiques par la France, il apparaît indispensable d'intégrer ces enjeux dans la stratégie et la programmation financière et opérationnelle.

de M. Longuet. Je voterai ces amendements, mais il faut aussi tenir compte des pays qui nous entourent, car la pollution ne s'arrête pas aux frontières

quels étaient les facteurs influant sur les émissions de polluants. Il y a en gros quatre familles d'émetteurs : l'industrie, les transports, le secteur résidentiel et l'agriculture.

dans « la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de l'attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, et de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique

Il vise à inscrire, parmi les objectifs de la programmation des infrastructures, l'amélioration de la mobilité quotidienne à l'intérieur des massifs, en fluidifiant le trafic routier, notamment dans les territoires transfrontaliers.

entre 1999 et 2009, en Belgique, la part modale du fluvial est passée de 10 % à 18 %. Pour se rapprocher de ce niveau de performance, il est nécessaire d'engager une politique ambitieuse et incitative de développement du transport fluvial.

des programmes d'investissements routiers très importants pour les territoires d'outre-mer. Je pense à la route du littoral, à La Réunion, qui doit être notre investissement routier le plus important-

vote. Je ne peux me satisfaire de cette réponse. Cela fait des années que j'entends l'expression de cette bonne volonté.

dans le cadre de la mise en place des programmes d'investissement prioritaires.

Ainsi, régénérer les petites lignes, les lignes du quotidien, permettrait de maximiser l'usage du réseau existant et d'améliorer la mobilité sans avoir besoin d'artificialiser de nouvelles surfaces pour la construction d'infrastructures. Nous proposons également, dans une logique de transition écologique, de renforcer les dessertes par les trains Intercités, de jour comme de nuit, notamment en zones rurales. Les habitants de zones rurales excentrées doivent pouvoir participer à la vie nationale sans être contraints dans leur mobilité par le coût de celle-ci. Ils doivent pouvoir bénéficier d'une offre de transport qui permette des déplacements aller-retour dans la journée, et ne pas être contraints à effectuer de fastidieux et dangereux trajets de nuit en voiture, s'ils ont la chance d'en posséder une. Il s'agit de pouvoir se rendre non seulement à Paris, mais aussi dans les autres régions françaises.

Je pense notamment au Paris-Briançon, indispensable au désenclavement des Hautes-Alpes. Il nous semble particulièrement opportun de faire référence au transport ferroviaire et au développement des dessertes par trains Intercités de jour et de nuit dans le présent article, tant ce mode de transport apporte d'avantages en termes de confort et de sécurité aux personnes, et d'avantages économiques et écologiques à notre pays.

de la commission ? Le doublement de la part du ferroviaire constitue un objectif du programme d'investissements prioritaires n° 2. Le rapport annexé prévoit « un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains

: La parole est à M. Éric Gold. Il est prématuré et limitatif de déterminer si l'objectif de désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales doit uniquement s'effectuer grâce à des aménagements existants.

vue du désenclavement d'une ville moyenne ou d'un territoire rural, les aménagements d'itinéraires existants ne peuvent pas apporter une véritable réponse. Des procédures comme la déclaration d'utilité publique, les acquisitions foncières ou les aménagements fonciers

Des travaux sont parfois attendus depuis plusieurs générations de contrats de plan État-région, selon des calendriers lointains. Il faut privilégier cet objectif plutôt que la construction de nouvelles infrastructures. 1 milliard d'euros sera consacré sur dix ans à l'amélioration de la qualité de la desserte de notre réseau routier national ; il s'agit d'opérations très concrètes, comme le précise le rapport annexé- déviations courtes, aménagements

Le programme d'investissement relatif au désenclavement routier doit permettre à l'État de consacrer de l'argent à la remise en état du réseau routier national. L'objectif d'équilibre territorial me semble tout à fait satisfait par l'alinéa 3, qui prévoit la réduction des inégalités territoriales.

: La parole est à M. Martin Lévrier. La rédaction actuelle de l'article met l'accent sur le développement de l'usage des mobilités propres et partagées. Dans une démarche de mise en place de l'innovation, il paraît cohérent de viser le développement des mobilités en général.

l'article 1 A du projet de loi d'orientation des mobilités prévoit la mise en place de cinq programmes d'investissements prioritaires. L'un de ceux-ci a trait au soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, notamment par le renforcement de l'accessibilité des ports et des grands itinéraires internationaux ferroviaires et fluviaux. Cet amendement vise à associer à une politique de transport ambitieuse le développement du transport propre par le déploiement de véhicules de transport des marchandises à faibles émissions. En effet, le maintien et le développement de la compétitivité des transports de marchandises peuvent se conjuguer avec le verdissement de ce secteur. Le déploiement de véhicules à faibles et très faibles émissions, fonctionnant à l'électricité, à l'hydrogène ou au bio GNV, permet d'assurer la décarbonation du transport de marchandises.

des dispositifs de soutien aux infrastructures de recharge, sachant que le texte prévoit une prise en charge par le gestionnaire de réseau d'une part plus importante des coûts de raccordement, ce qui conduira à une division par deux

en mission, les constats demeurent les mêmes : urgence écologique, nécessité d'un changement de paradigme, maîtrise des externalités négatives du transport de marchandises, pertinence du fret ferroviaire ... La liste n'est pas exhaustive. Ainsi, du Grenelle de l'environnement à la COP 21, tout le monde a pieusement approuvé certaines recommandations, par exemple assurer le maillage du territoire et développer le fret ferroviaire pour contenir le trafic de poids lourds, mais voilà vingt ans que le réseau ferroviaire se transforme à rebours de ces directives. Les fermetures de services, de lignes, de gares de triage continuent, de même que les cessions de matériel roulant. Les 3 200 kilomètres de réseau secondaire sont encore en danger d'abandon pur et simple, faute d'investissements. Que veut dire l'expression « maintien du fret ferroviaire là où il est pertinent »

? Pourtant, les rapports sur les décès dus à la pollution de l'air se multiplient. Pourtant, l'urgence climatique n'a jamais été aussi forte. Il est dès lors irresponsable de penser les transports de demain

Ce réseau est indispensable au développement du fret de proximité, puisqu'il permet d'accomplir le dernier kilomètre et de limiter les transferts d'un moyen de locomotion à un autre. Ce dont la France a besoin, c'est d'une grande politique publique de transport de marchandises, qui doit reposer sur un réseau ferré au maillage fin permettant d'irriguer les territoires tout en répondant aux besoins des entreprises et des citoyens. Très bien ! Quel est l'avis

25 % des marchandises transportées passent par des lignes capillaires. De fait, il y a déjà un soutien de l'État à la remise en état de ces lignes capillaires, à hauteur de 10 millions d'euros par an, l'Afitf. Par ailleurs, nous soutenons le développement

Bérit-Débat. Au travers de cet amendement, nous proposons que l'État lève un emprunt à moyen et long terme afin de financer les investissements dans les infrastructures prévus par le projet de loi.

puisqu'il manquera 500 millions d'euros par an à l'Afitf à partir de 2020. La commission du développement durable du Sénat a dû sanctuariser l'affectation à l'Afitf du produit de l'augmentation de la TICPE prévue par la loi de finances pour 2015. Malgré

à n'y rien comprendre ! Plusieurs raisons militent donc en faveur de la levée d'un emprunt à long terme pour financer les infrastructures dans un contexte particulièrement difficile, sur fond de crise des « gilets jaunes » et de montée de l'intolérance à l'impôt.

Tous les indicateurs sont aujourd'hui au vert. Selon la Banque de France, la charge de la dette devrait baisser, en 2021, de près de 10 milliards d'euros. Notre amendement s'inscrit bien dans une logique de « déficit sans pleurs

C'est précisément dans ce contexte de ralentissement que l'on observe, aux dires de certains économistes, que les mesures prises pour répondre à la crise des « gilets jaunes » auraient permis un léger effet de relance de l'économie. Il faut continuer dans cette voie. Il est particulièrement utile, dans une conjoncture de croissance atone,

au défi du réchauffement climatique : comment ne pas évoquer des mécanismes simples et sains, que de très nombreux pays ont mis

On regardera sans doute demain comme un grand paradoxe que, par manque de crédibilité et de confiance mutuelle, des États qui empruntaient à 0,7 % dans un contexte de croissance nominale de 3 % n'aient pas davantage tiré parti d'une fenêtre aussi exceptionnelle. La dette publique française frôle aujourd'hui 100 % du produit intérieur brut du pays. Il est inévitable et salutaire que l'approche de ce seuil suscite un débat. Sommes-nous en danger ? Quelles stratégies adopter pour réduire la dette ? Commençons par l'évidence : il n'y a pas de risque immédiat. Nous sommes toujours dans une période de déficits sans pleurs parce que l'État français emprunte sur dix ans à un taux nettement inférieur à 1 %, qui ne compense même pas l'inflation. Tendanciellement, si cela continue, la charge des intérêts représentera moins de 1 point de PIB, comme à la fin des années 1970, lorsque la dette ne pesait que 20 % du PIB. les taux vont remonter, mais sans doute lentement et, surtout, la maturité moyenne de la dette est de plus de sept ans. Quand bien même la normalisation serait brutale, l'impact sur la charge annuelle d'intérêts demeurera graduel. » Merci à Jean Pisani-Ferry

Ces contrats qui lient l'État aux établissements publics cités sont conclus pour dix ans et réactualisés tous les trois ans. De fait,

pour en finir avec l'avantage concurrentiel déloyal dont bénéficie la route par rapport au rail pour le transport de marchandises. Comment réorienter le transit vers les voies de transport les plus vertueuses écologiquement si les usagers de la route continuent de ne pas financer les infrastructures, contrairement à ceux des autres modes de transport ? Il s'agit simplement, conformément au droit européen, de mettre en place une fiscalité juste socialement et écologiquement, une fiscalité qui nous semble bien plus juste que l'augmentation des prix à la pompe et de la TICPE. Le précédent gouvernement, empêtré dans un montage juridique et financier intenable, avait reculé, mais nous considérons que la question est toujours posée

qui leur sont adossés reste limitée et lacunaire. En particulier, le troisième des cinq programmes d'investissement prioritaire restreint la problématique du désenclavement des villes moyennes et des régions rurales à un désenclavement routier, ce qui ne nous semble pas satisfaisant. Nous proposons donc de parler de désenclavement routier et ferroviaire, puisque le désenclavement des territoires passe également par le rail à nos yeux. Certes, cette question est en partie traitée au travers du deuxième programme, qui concerne les noeuds ferroviaires, mais nous estimons qu'il est nécessaire d'y faire référence explicitement à propos de l'enjeu du désenclavement. Nous pensons en effet que, pour lutter contre les fractures territoriales, il est essentiel de régénérer les « petites lignes », les lignes du quotidien, et de permettre ainsi de maximiser l'usage du réseau existant pour améliorer la mobilité sans artificialiser de nouvelles surfaces par la construction d'infrastructures.

la référence à la montagne figurant dans la rédaction des alinéas 18 et 44 trouve sa justification dans la spécificité « montagne » reconnue par la loi modifiée n° 85-30 du 9 janvier 1985. L'indication, à l'alinéa 32, que l'État reprendra une politique d'investissement dans les trains d'équilibre du territoire et les deux trains d'aménagement du territoire- les trains de nuit Paris-Briançon et Paris-Rodez -permet d'envisager la possibilité de mettre en place d'autres trains de nuit sur de nouvelles liaisons, pour desservir les Pyrénées, par exemple, et, pourquoi pas, le coeur du Massif central. Aurillac était desservie par un train de nuit qui a été supprimé en 2013. Cela a contribué à aggraver encore, de façon très importante, Enfin, le complément rédactionnel, à l'alinéa 47, a pour objet de rappeler que les travaux d'entretien, de sécurisation et de modernisation du réseau routier national concernent également d'importants ouvrages de prévention des risques naturels, particulièrement nécessaires en zone de montagne.

Merci